Bonsoir mes chers collègues, Madame la Ministre, la séance est reprise, nous reprenons donc la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 768 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l'article 15. Qui prend la parole pour l'amendement 768 Monsieur Dantec. Merci madame la la présidente, le rapport annuel banking Carlos publié en mars dernier, révèle que les banques françaises en financer les énergies fossiles pour 230 3 20 15 milliards de dollars depuis l'adoption des accords de Paris pour le climat, d'après cette estimation, elles ont même dépassé leurs voisines britanniques illustrant un écart croissant entre les promesses de finance verte de la place de Paris et les pratiques réelles sur le climat. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que nous ne pouvons parvenir à l'objectif de neutralité carbone pour 2050 si le secteur financier ne connaît pas lui-même l'impact de ces investissements sur le climat en avril dernier, je le souligne, la Nouvelle-Zélande devenait le 1er pays au monde à exiger de ses mangues, la transparence des impacts écologiques des investissements réalisés, certains pourraient peut-être penser que le le sens de cet amendement et de stigmatiser les banques françaises, pas du tout. Les banques françaises ont aujourd'hui des stratégies assez différentes, je n'en citerai évidemment aucune certaines n'ont pas changé leur stratégie d'investissement, d'autres les ont modifié et y compris les ONG essaye aujourd'hui de faire la la différence entre les réalités des stratégies des unes et des autres à court et moyen terme donc, cet amendement vise à exiger des banques d'adjoindre à leur bilan annuel de compte un état des lieux des émissions de carbone générées par leurs investissements dans chaque pays et pousser ainsi la France à devenir un pays beaucoup plus transparent, c'est un enjeu majeur pour la place de Paris, il y a eu au moment j'en étais un des spectateurs au moment de, de la à Paris des engagements assez fort de la place parisienne non dénué d'ailleurs d'arrière-pensées dans le cadre d'une compétition qu'on connaît avec un la City à Londres et il est évident, demain, que la place financière qui va s'imposer sera celle qui sera la plus transparente sur les questions climatiques donc derrière cet amendement, il y a effectivement la nécessité de mettre les banques devant leurs responsabilités, lui aussi, derrière cette transparence et la capacité de faire la différence entre celles qui sont en évolution et celles qui ne veulent pas évoluer la possibilité, l'opportunité de renforcer la place de Paris et je crois que cet amendement devrait donc largement consensuel. Si cher collègue, monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît. Madame la présente, Madame la Ministre, cet amendement 700 longs 68 rectifié porte sur un Champ très large d'entreprise. il pourrait, par ailleurs, il pourrait, pardon, par ailleurs, conduire à la révélation données sensibles pour notre secteur bancaire national en outre juridiquement il s'insère dans un article du Code monétaire et financier traitant des pays non coopératifs et cela n'est pas forcément très adapté pour ces raisons de forme et de fond, c'est une demande de retrait. Et à défaut, un avis défavorable, chers collègues. Merci, monsieur le rapporteur, Madame la Ministre votre avis. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, ravi de vous retrouver sur l'examen de ce texte, alors, Monsieur le Sénateur, Dantec effectivement sur cette demande d'obligation de publication du bilan des émissions de gaz à effet de serre, je partage évidemment pleinement vos intentions, vous le savez, d'ailleurs, elles font écho à une action récente du gouvernement dans le décret d'application de l'article 29 de la loi énergie-climat qui est venu modifier l'article L. 533 22 1 du Code monétaire et financier, en prenant en compte donc dans la politique d'investissement, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et les moyens mis en oeuvre par les les investisseurs pour contribuer à la transition, nous avons également effectivement au niveau européen des acteurs financiers qui sont soumis à des obligations de transparence concernant la durabilité de leur investissement au titre des règlements du paquet finance durable de 2000 19 et ces textes, ils permettront aux parties prenantes d'identifier avec précision les actions des acteurs financière la matière, notamment sur la décarbonation de leur portefeuille j'estime donc effectivement que les dispositions actuellement en vigueur, répondent aux préoccupations que vous soulevez, c'est donc une demande de retrait sinon avis défavorable. Monsieur Dantec je mets aux voix vous retirer en mai aux voix, alors avec 2 avis défavorables qui vote pour.

Qui vote contre. Alors on va faire un assis debout parce qu'on a, vous êtes à égalité, désolé, il y a, il y a mais qui sont arrivés en entre-temps allez un assis debout alors écoutez, c'est la présidente qui décide, je vous demande de faire un assis de qui pour.

19 19 vous avez pu recompter comme moi, donc il n'est pas adopté l'amendement 791. L'amendement 791 et défendu.

Cet amendement vise à flécher prioritairement à l'action de la banque publique d'investissement, la BPI vers la transition écologique, il permet ainsi de s'assurer que les projets bénéficiant de fonds publics soient en adéquation avec les enjeux environnementaux. Oleg est efficace, monsieur le rapporteur. Si madame la présidente, il me semble pertinent de mettre à jour le texte fondateur de la banque publique d'investissement pour y inscrire la transformation sociale et écologique des entreprises françaises ce titre agi d'un avis favorable. Merci, monsieur le rapporteur, Madame la Ministre votre avis aurait générerait ou non un impact social ou écologique positif est une tâche sans doute complet. Délicate à a qualifié par ailleurs des pays s'est déjà dotée d'un plan climat qui est doté de 20 milliards pour accélérer la transition écologique des entreprises, c'est donc un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre, je mets donc aux voix cet amendement avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui vote pour. Contre qui s'abstient-il être adopté, nous avons maintenant 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 810 Monsieur Gay. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je suis certain que Madame la Ministre, sera d'accord avec cet amendement, puisqu'il s'agit d'un cours de la part des investissements durables sur le plan environnemental de la Caisse des dépôts. Il y a évidemment une volonté politique très forte du gouvernement d'appliquer l'accord de Paris et de faire beaucoup de choses en matière environnementale, sur le plan international et donc du coup nous pensons simplement qu'il serait juste que les outils publics à sa disposition, soit en adéquation avec cette politique tellement forte menée sur le plan environnemental. Pour le coup, nous notons une. Nous notons une avancée puisque le 29 octobre dernier le groupe Caisse des dépôts, a annoncé le renforcement de l'encadrement de ce financement aux énergies fossiles. C'est une première avancée, mais nous pensons que nous pouvons aller plus loin, par exemple, l'ONG Oxfam a dit qu'encore 10 euros prêtés par les banques françaises n'autre pas mon par la Caisse des dépôts, cette aller aux énergies fossiles, contre 3 seulement aux énergies renouvelables, donc, pour le coup. Il y a les banques privées qui font plus un peu plus même que la Caisse des dépôts sur cette question-là, et il apparaît on ne comprendrait pas pourquoi on n'adopterait pas ce cet amendement parce que la Caisse des dépôts, doit être en première ligne sur les investissements d'avenir et sur le plan environnemental et, par exemple, d'arrêter de financer le tout charbon vous voyez parce qu'on ne peut avoir le débat l'an dernier pour arrêter les centrales à charbon sur notre territoire et on ne comprendrait pas pourquoi elle continuerait à le financer ailleurs dans le monde à travers aux entreprises françaises, donc c'est simplement carrément même un amendement de coordination que nous vous proposons. Merci, cher collègue, l'amendement 792 Monsieur Dantec. Oui, donc autre amendement rédactionnel qui va dans le même sens, mais bon, même si nous commençons avec beaucoup de sourires, c'est quand même un sujet important, la, la Caisse des dépôts et un des acteurs majeurs de la transition énergétique et de la capacité de la France à tenir l'objectif de moins 55 % que nous avons mis en chapeau de de ce texte et donc, nous vous proposons un alinéa très clair qui est, ces investissements sont conditionnés à la publication par les entreprises de plan de transition alignés avec les grands objectifs climatiques fixés au niveau national, en particulier le plafond national des émissions de gaz à effet de serre définis par grands secteurs, les entreprises vont le faire. Il est clair aujourd'hui, ne serait-ce que par la pression des actionnaires que toutes les grandes entreprises vont devoir ou le fonds des gens pour un certain nombre d'entre elles présenté leur stratégie sous un angle de neutralité carbone et un climat de Friendly, comme on dit en bon français, donc que la Caisse des dépôts, aille dans ce sens-là et ne finance que des entreprises qui respectent les objectifs nationaux et, globalement, la part de la responsabilité je crois que c'est de de bonne politique je rajouterais aussi madame la la ministre, que c'est l'occasion d'insister sur le fait que la Caisse des dépôts et la banque des territoires est un acteur majeur de la capacité de nos collectivités là aussi à investir plus rapidement qu'il faudra même peut-être même si ça n'est pas dans le cas de ce projet de loi prévoir demain des Budgets annexes des collectivités territoriales pour leur effort énergétique et bien distinguer l'investissement classique qui augmente, les services aux habitants des investissements notamment qui amène derrière plutôt à à des baisses de, de coûts de fonctionnement et qu'aujourd'hui dans nos Budgets d'investissement ne distingue pas les 2 et que ça pose des des problèmes de visibilité de la réalité de l'investissement et de l'endettement des des collectivités territoriales, tout ça pour dire que, avec la Caisse des dépôts, on a un acteur majeur cet acteur majeur doit être aligné sur l'ambition que le Sénat, de manière quasi unanime a rappelé en introduction de ce projet de loi. Merci, cher collègue, pour ces explications d'amendement de coordination, monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente, sur l'amendement 810 toute façon particulièrement synthétique le la conditionnalité environnementale des financements de la Caisse des dépôts pourrait limiter les capacités de financement de l'économie française, notamment des PME, à ce titre, la commission émet un avis défavorable. Concernant l'amendement 792 la conditionnalité des financements de la Caisse des dépôts à la publication par les entreprises de plan de transition alignés avec les grands objectifs climatiques fixés au niveau national et particulièrement lourde et pour limiter les capacités de financement de l'économie française, notamment des PME, également en avis défavorable qui est proposé. Merci, monsieur le rapporteur, Madame la ministre. sur la volonté à nouveau un d'encourager le financement dans la transition écologique bien sûr nous nous partageons ce souhait et d'ailleurs nous nous le mettons en oeuvre dans le plan de relance, on va le voir, mais techniquement d'abord, il semble difficile d'analyser, voire impossible même d'analyser tout le stock de de prêts aux PME pour savoir si ce financement contribue à des activités durables, d'autant que les lignes de prêts PME ne finance pas nécessairement un projet ciblé la Commission européenne a, somme toute, entendu à cette difficulté et va concevoir l'élaboration de lignes directrices spécifiques pour le calcul des ratios d'alignement des bilans bancaires sur la future taxonomie durable européenne dans le plan de relance donc qui prévoit un plusieurs mesures beaucoup plus concrètes. Pour financer la transition 105 millions d'euros de crédits d'impôts pour les investissements de rénovation des bâtiments par exemple des TPE et PME dans le secteur tertiaire 15 millions pour l'accélération de la transition de 45000 artisans commerçants et indépendants ou 35 millions pour la mise à disposition d'aide forfaitaire pour les actions et investissements dans l'éco-conception de produits et on pourrait également parler des 45 millions pour la mise en place d'actions d'accompagnement des entreprises engagées dans la transition, nous avons là des des leviers concrets et immédiatement mobilisables opérationnel, c'est donc sur le 810 un avis défavorable concernant l'amendement 792 défendu par le sénateur Dantec ici donc, cet amendement, il se concentre sur les entreprises sur le financement des entreprises n'est qu'une des activités de la CDC et remplacer la notion de développement durable par la transition écologique et énergétique des entreprises reviendrait ainsi à adopter une vision restrictive du Champ d'action avec effectivement une CDC qui est déjà très engagée dans une politique d'investissement écologique volontariste et qui fait l'objet d'ailleurs d'un bilan annuel et qui obtient de très bons résultats, c'est donc un avis défavorable. Merci madame la ministre, monsieur Dantec, vous avez demandé la parole pour expliquer. Je je je suis assez insatisfait, je dois l'avouer des réponses apportées. Les émissions françaises la déclinaison de l'objectif européen de moins 55 % ce sont globalement les émissions cadastrale

bras financier de l'État va de moins financer des entreprises qui pourraient réaugmenter les émissions françaises en contradiction avec l'objectif de moins 55 % ça n'est en fait pas possible monsieur le rapporteur, comment peut-on dire que ça pourrait être pénalisé l'économie française, alors que derrière, c'est clairement le cadre économique, y compris de régulation avec des taxes aux frontières sur le le CO2 émis par des pays qui serait moins ambitieux, qui est l'enjeu, c'est une contradiction flagrante, c'est une contradiction flagrante, moi je, je reste convaincu et vous m'entendrez encore le dire dans les 15 prochains jours que tout l'enjeu de ce projet de loi, c'est la mise en cohérence de l'ensemble de nos bras d'intervention sur l'économie et sur la vie quotidienne des Français, et là, votre réponse va toujours dans le sens et c'est aussi un peu le sens de la réponse de Madame la Ministre, de dire on fait du climat, de manière un peu périphérique on va soutenir ce qui ce qui avance, mais on ne va pas au coeur de nos leviers, or la Caisse des dépôts et le coeur, un des coeurs de levier de notre capacité à faire avancer l'économie française, par ailleurs, et nous sommes tous d'accord là-dessus, on est dans une logique, et y compris la taxe carbone aux frontières doit aller dans ce sens-là, avec des impacts très positifs sur l'emploi, sur le fait de dire que nous allons protéger l'économie européenne des des pays qui ne respectent pas les, les, les contraintes d'émission mais que donc, sinon on rerentre des entreprises sans regarder si elle-même en ramenant les procès sur le territoire national, européen, ne respectent pas, ce cadre d'émission en fait, on remet en en difficulté tout le cadre international qui a permis de rentrer les entreprises et je pense qu'on est vraiment, et c'est très sincère, ce que je dis dans un moment où on n'arrive pas à créer une cohérence d'ensemble et je pense que, effectivement, la Caisse des dépôts, que ce soit son action sur les collectivités territoriales, avec la banque des territoires ou sur des entreprises importantes française doit être au coeur et je trouve que là on a des réponses qui laisse finalement nos grands leviers en périphérie de l'effort climatique. Si cher collègue Monsieur Gay, vous avez demandé la parole, explications de vote également. Merci madame la présidente, oui, moi aussi je suis ne satisfait des réponses apportées et par monsieur le rapporteur, et pardon, Madame la Ministre, ce que j'ai toujours un peu de mal à comprendre. Lorsque les gens doivent faire valoir leurs droits en France droit au chômage, droits à la retraite, droits sur un accident du travail, là il y a pas de problème, on contrôle et on contrôle même strictement normal. Mais lorsqu'on parle d'argent public d'honneur de entreprises ou de l'argent public donné à travers une banque publique pour aider un financement, alors là, quand on vous parle de contrôle ou de conditionnalité tout devient impossible, c'est pas possible, on va pénaliser les entreprises, c'est pas possible, c'est pas le droit européen, c'est pas possible, vous imaginez qu'est ce qu'on ferait, et donc là vous avez une petite contradiction, y compris moi, je pense que le dans le débat, où nous en sommes. Sur de l'argent prêté à des entreprises, la sur la question environnementale ou en maintien de l'emploi et de sites industriels, on devrait dire aux entreprises et la Caisse des dépôts pourrait être la première c'est du gagnant-gagnant on va accompagner l'entreprise, on vous prête de l'argent public sur un projet, on l'étudie, avec vous on mais avec vous, un comité d'experts pour vous accompagner, y compris vers la transition écologique. Et puis on fait un point chaque année si on avance, on continue, mais si on voit que l'argent public n'a pas été. Bien utilisé sur la transition. énergétique écologique ah ben on arrête. Voir on sanctionne, mais là, je sais que c'est un grand mot pour vous et donc j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi nous sommes en incapacité de créer des mécanismes pour conditionner les aides publiques ou les prêts publics, y compris à travers la Caisse des dépôts, faudra bien m'expliquer pourquoi il y a ce blocage, je vous remercie.

Oui, madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je présente cet amendement porté par notre collègue Didier Marie, compte tenu des difficultés exceptionnelles d'exécution des contrats provoquée par la crise sanitaire, l'état d'urgence sanitaire a permis d'assouplir les conditions de passation des marchés publics, l'objectif était double : lutter contre le gaspillage alimentaire et si vous regardez les emplois en soutenant en particulier les producteurs agricoles dont l'activité a été fortement impactés par les mesures prises pour limiter l'épidémie le présent amendement vise donc à pérenniser cette assouplissement des conditions de passation de marchés publics pour les fournitures, de denrées alimentaires enfin durablement soutenir notre production agricole et alimentaire locale. Merci, chers collègue Madame la rapporteure votre avis s'il vous plaît. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, alors il s'agit donc d'une demande de de pérennisation de l'assouplissement des conditions de passagers passation des marchés publics pour les denrées alimentaires, mon cher collègue, nous ne pouvons malheureusement pas pérenniser la dérogation conjoncturel qui qui fait l'objet de cet article, au-delà de la durée qui est précisé puisque le faire nous mettrait risque à nous mettre en non conformité avec à la fois notre droit constitutionnel et le droit européen pour des principes d'égalité de traitement de libre accès à la commande publique ou de non-discrimination qui ont été largement évoqués au cours de cette séance, donc un avis défavorable. Merci madame la ministre. ministre. également un avis défavorable pour les raisons précédemment évoqués par Madame la rapporteure avec une dérogation au principe de la commande publique qui n'a été autorisée par le Conseil d'État, que dans le cadre d'une mesure d'intérêt général mais temporaire lié à la situation d'urgence que nous savons, et donc sur une période donnée, c'est donc un avis défavorable. Merci madame la ministre, je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui tour. Abstention

après la fin de l'état d'urgence sanitaire, il sera possible de conclure des marchés publics, agroalimentaire, dès lors qu'ils seront inférieurs à 100000 euros hors taxes sans publicité ni mise en concurrence préalable. Cet article je le partage, je partage son objectif, il introduit une souplesse qui peut aider le secteur agricole qui, parfois, été dans certains domaines impactés par la crise et la fermeture des débouchés l'article précise que les acheteurs devront veiller à choisir une offre pertinente mon amendement précise que l'pertinente doit prendre en compte la lutte contre le gaspillage alimentaire l'impact environnemental et les retombées attendues en termes d'emploi local ils renforcent donc la portée de cet article. Merci, cher collègue Madame la rapporteure. C'est un amendement qui vient compléter judicieusement l'appréciation de la pertinence et donc un avis favorable. Merci madame la ministre, ma vie. Il me semble que malheureusement cette cette disposition qui a été prise, elle nous permet d'assurer une certaine réactivité, une conclusion rapide des marchés publics de denrées alimentaires, notamment pour limiter la durée de de stockage des denrées qui peuvent être périssable, le principe était donc vraiment la plus grande souplesse et la réactivité et ajouter des contraintes supplémentaires aux acheteurs pourrait freiner cette cette mesure et ça et sa mise en oeuvre rapide et donc en limiter considérablement le bénéfice est donc un avis défavorable. Merci, je mets donc aux voix cet amendement avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui vote pour.

nous avons maintenant des amendements sur l'article additionnel, le 5 amendements identiques le 41, défendu par Monsieur Madame la présidente, mes chers collègues, donc cet amendement se veut complémentaire de la loi Egalim mais l'améliorer, il vise à valoriser les produits de circuits de proximité locaux à faible coût environnemental en dérogeant à titre expérimental pour un certain pourcentage de denrées au principe d'égalité de traitement des candidats prévue à l'Arctique L 3 du code de commandes publiques, dans le but donc de soutenir l'ensemble des acteurs du système alimentaire locale et de contribuer au développement économique et social des territoires merci. Merci, cher collègue, le 69 n'est pas défendu le CIV Monsieur 2000. Oui merci madame la présidente, la loi dite Egalim de 2018 à instaurer des objectifs ambitieux en matière d'approvisionnement de la restauration collective, pour autant, il est important que la liste des produits éligibles au 50 % de produits durables de qualité au sens de la loi Egalim bénéficie aux denrées alimentaires produites sur les territoires de proximité et vertueuse, d'un point de vue environnemental, je pense en particulier à la saisonnalité, je pense à la fraîcheur où je pense encore le risque observée aujourd'hui pour en avoir discuté avec de nombreux professionnels de la restauration collective et que ces mesures encouragent l'achat de produits peu ou moins vertueux en termes de conditions de production et d'exigence de qualité pour le reste des approvisionnements car les produits durables et de qualité, présente un coût généralement plus élevé le présent amendement se veut donc complémentaires des objectifs fixés par la loi Egalim il vise à valoriser les produits issus de circuits de proximité locaux et à faible coût environnemental en dérogeant à titre expérimental et pour un certain pourcentage de denrées au principe d'égalité de traitement des candidats prévue par le droit de la commande publique, l'introduction de produits alimentaires de proximité permettrait bien sûr, vous l'avez compris de soutenir l'ensemble des acteurs du système alimentaire locale est ainsi bien sûr, de contribuer au développement économique et social de nos territoires. Merci, cher collègue, l'amendement 111 monsieur Delcros. Il est défendu très bien, merci le 1780 n'est pas défendu madame le rapporteur, votre avis sur ces

qui est de mieux valoriser les produits locaux et quasi satisfaite en fait par le texte que la commission vous proposera à l'article 60 articles dans lequel nous avons essayé de mieux intégrer les produits locaux issus de circuits courts, ainsi que les produits issus des plans alimentaires territoriaux dans les approvisionnements en restauration collective en essayant de faire en sorte qu'une fois plus, plus conforme possible à la fois au droit constitutionnel ou au droit européen, par ailleurs, donc, et cela a déjà été évoqué ce type d'argument et est contraire au droit constitutionnel au droit de l'Union européenne, puisque je le rappelle, hein, il s'oppose à la prise en compte en tant que critère explicitement affiché dérogatoire d'un critère de préférence géographique dans l'attribution des marchés, cela dit, je pense que vous aurez à coeur, Madame la Ministre, peut-être, de rebondir sur ce sujet majeur pour pour nos nos territoires, la prise en compte des, des, des produits locaux de proximité et peut-être que lors de la présidence à venir de la France dans l'Union européenne en janvier 2022 c'est une une disposition que vous pourriez apporter, elle a d'ailleurs donc été préconisée dans le cas du groupe de travail alimentation durable et locale que notre commission des affaires économiques à mener la commission du développement durable et puis pour assurer un peu mes, mes collègues, je dirais qu'il existe quand même aujourd'hui un certain nombre de pratiques que connaissent bien les gestionnaires ou nos agents dans les collectivités, qui consiste en fait à à mettre des spécificités fication technique des priorités sur un certain nombre de produits de qualité sous Label et qui permet en fait d'atteindre ses objectifs de produits locaux et puis enfin un guide des clauses à inclure dans les marchés publics a été publié donc dans ce sens, d'accompagnement des des gestionnaires, il y a 2 mois par le Conseil national de la restauration collective. Merci, cher collègue, madame la ministre. nous le partageons ce ce besoin de promouvoir les produits locaux, et d'ailleurs nous avons beaucoup oeuvré ensemble à ce ce levier ce renforcement de la souveraineté alimentaire, c'est tout l'article 15 bis que vous venez de d'adopter, je crois qu'on peut s'en féliciter, seulement, effectivement, vous le savez, il n'est pas possible de faire référence, même à titre expérimental à ce ce critère géographique hein de de localisme dans la passation de marchés publics, c'est un principe du droit de la commande publique et c'est également effectivement un enjeu de compatibilité européenne que le gouvernement et je je m'y engage, madame le rapport. Portera fortement au plan européen pour plaider en faveur d'une plus grande souplesse dans les approvisionnements alimentaires de proximité en cette attente, je vous propose que nous restions exemplaire en la matière. Merci madame la ministre, à Monsieur Chassaing monsieur Demilly Monsieur Delcros est-ce que vous retirez l'amendement suite à la demande de la commission.

Merci madame la présidente, madame la Ministre pour vous redire notre mécontentement, vous le savez, sur le fait que le Sénat ne puisse pas se prononcer sur le s'étant d'ailleurs, il y a un peu plus de 2 mois, ici même, notre groupe avait déposé une proposition de résolution adoptée à l'unanimité moins quelques abstentions et je le reconnais, nous avions eu un débat d'extrême qualité où chacun et chacune des groupes a pu s'exprimer et je vais le dire comme ça je encore mais sensibilités a a dit un certain nombre de réserves. Sur l'opportunité de prolonger le s'étend, mais en tout cas nous avons toutes et tous, dit que nous voulions Lyon au revoir le débat. Pour l'instant, nous sommes empêchés. Très bien, et le président de la République a répété il y a peu. Si. Je un rapport qui me dit que le CETA va à l'encontre des accords de Paris alors j'envisagerais un moratoire et la Convention citoyenne a redit qu'elle souhaitait pour sa part, les 150 citoyens plutôt un moratoire sur l'ensemble des traités de libre-échange, et particulièrement le s'étale Marco alors nous ben nous y disons chiche au président de la République, puisque nous sommes empêchés d'débattre, nous vous proposons de faire un moratoire sur l'opportunité d'un moratoire sur ce traité de libre-échange au moins nous aurons les données et puis bah, comme ça nous pourrons si c'est le cas et si ce ce rapport que vous pourrez pas nous que vous Ferez monde que cet accord va à l'encontre des accords de Paris, peut-être que le président de la République pourra envisager potentiellement un moratoire voilà donc j'espère au minimum. Que nous allons pouvoir au moins avoir un petit débat et peut-être l'opportunité de le voter collectivement, chacun et chacune le président Jean rien de ce qu'il pense du 7 nous demandons bien un rapport sur l'opportunité ou pas de moratoire. Si ce cet art et cet accord de libre-échange. Contrevient ou non aux accords de Paris voilà et je pense que c'est une pièce de plus mis dans la volonté, entendait bien, Madame la Ministre, que nous ayons en finalement ce débat ici dans l'hémicycle, je vous remercie. Merci, chers Madame la rapporteure votre avis. Merci madame la présidente, donc je pense que nous l'avons tous compris, il s'agit d'un amendement d'appel pour pour rebondir sur ce sujet qui tient à coeur à notre collègue et qui nous tient tous d'ailleurs à coeur puisque nous souhaiterions effectivement pouvoir débattre sur ce sujet du CETA. Donc ce sera un avis plutôt défavorable sur sur ce rapport de moratoire, mais je pense que nous attendons tous avec impatience les les propos de Madame la ministre. Madame la ministre, donc. hein, vous le vous le savez, nous avons tenu à mettre les les alertes et même les freins nécessaires à la la ratification de du et au respect de l'accord de Paris dans tout accord d'ailleurs commercial aujourd'hui, nous avons tous ce souci il est largement partagée d'ailleurs sous l'impulsion de la France, cette ambition, elle a été inscrite dans le pacte Vert le Green Dean et dans la stratégie commerciale de la Commission européenne, donc je crois que aujourd'hui les lignes rouges ont été clairement fixé la France s'en est largement le travail, le travail sur ces questions, la réflexion, le débat doit évidemment se poursuivre pour préfigurer les les futurs A des futurs accords bien évidemment et je crois d'ailleurs que les parlementaires ont tout loisir de se saisir de tout sujet qui c'est sur le format effectivement sur le format du rapport, c'est un avis défavorable. Merci madame la ministre, je mets donc aux voix cet amendement numéro 143 avec un avis plutôt défavorable de la commission est défavorable du gouvernement qui vote pour. Qui vote contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté. Nous avons à présent 2 amendements identiques à l'article 15 ter le 64 Madame Di Folco. Merci madame la présidente, il s'agit de supprimer la disposition qui impose à l'acheteur public pour la rénovation et la construction de bâtiments, le recours à 25 % des matériaux biosourcés sourcées ou à bas carbone la décarbonisation ne saurait constituer un objectif atteignable avec le bio-sourcées le GO sourcées ou le bas carbone une ambition environnement environnementales national doit mobiliser les atouts et les expertises de l'ensemble des matériaux et des filières partageant les objectifs de diminution de l'empreinte carbone, les industriels des matériaux de construction se sont déjà saisis de ces enjeux avec des engagements volontariste de baisse de leur propres empreintes donc le choix fait en faveur de ces matériaux repose sur des postulats environnementaux biaisé, d'où la demande de suppression de cet article, merci.

cette suppression n'a pas lieu d'être, car la commission des affaires économiques, a veillé encadrer les effets de bord de cet article, d'abord en limitant aux constructions à l'exclusion des rénovations en deuxièmement en mettant les matériaux Géo sur c'est et bas carbone sur le même plan que ce bio-sourcées supprimant donc toute distorsion donc concurrence entre les différentes filières, des matériaux de construction et en prévoyant une date d'application au 1er janvier 2030 dans un sens plus conforme à la réglementation environnementale et romarin ce bornage travailler en amont avec l'ensemble des acteurs est équilibré, donc c'est une demande de retrait ou sinon un avis défavorable sur cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur, Madame la Ministre votre avis s'il vous plaît. cette obligation d'incorporation de matériaux biosourcés dans un quart de rénovation et de construction dans le dans lesquels intervient la commande publique, l'Assemblée nationale l'adopté avec un article qui qui la crée la commission du Sénat la limité la portée de cet article aux seuls travaux de de construction élargi aux matériaux éligibles aux matériaux Géo sur c'est au bas carbone, or le le gouvernement souhaite rétablir l'arrêt de la rédaction de l'article 15 ter, issue de l'assemblée pour viser la rénovation qui constituent un marché économique important pour les filières concernées et un domaine d'emploi également important pour la commande publique, cette commande publique, elle constitue un levier stratégique, hein, vous le savez, pour soutenir la croissance économique des filières de construction biosourcés je soutiendrai donc tout à l'heure, un amendement qui vise à revenir à la rédaction initiale votée par l'Assemblée, c'est donc un avis défavorable. Merci madame la ministre, je mets donc aux voix cet artiste cet amendement madame Di Folco.

l'atteinte des objectifs environnementaux pour répondre à l'urgence climatique nécessite d'engager une mobilisation massive et pérenne de l'ensemble des composantes du pays alors que les marchés publics de fourniture d'énergie pourrait constituer un levier stratégique pour la transition environnementale, pour l'instant, les dispositions de la commande publique en vigueur ne permettent pas aux acheteurs, il est temps, soumis de contribuer au déploiement des énergies renouvelables et donc à la transition écologique, il s'agit donc de lever des freins au progrès possibles dans le déploiement des énergies renouvelables aujourd'hui le droit de la commande publique, ne leur permet pas de s'engager dans le temps, lorsqu'il s'agit de fournitures courantes contraints d'acheter de telles fournitures sur une durée moyenne de 4 ans par la nécessité d'une remise en concurrence périodiques telle qu'interprétée par la jurisprudence ces acheteurs n'ont pas la possibilité de permettre aux opérateurs économiques d'amortir dans le temps une infrastructure nécessaire à la fourniture ou d'exiger que leur énergie soit produite par une nouvelle installation de production d'énergie renouvelable, ces acheteurs sont pourtant aujourd'hui nombreux à souhaiter faire preuve d'exemplarité en encourageant l'additionne IT, c'est-à-dire le développement d'installations de production d'énergie renouvelable, pouvoir mettre en oeuvre sur leur territoire les objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables, pouvoir programmer leur politique énergétique à plus ou moins long terme afin de maîtriser leurs coûts et leurs voulu cette disposition pourrait contribuer à l'atteinte des objectifs environnementaux, elle permettrait à l'État de se mettre en conformité avec le droit européen qui dit que les États membres et évalue les barrières administratives et réglementaires au contrat d'achat de long terme d'électricité renouvelable et supprime les barrières injustifiées et facilite le recours à de tels accords, je vous remercie. Merci, cher collègue, le 1200 ce monsieur 2. Merci madame la présidente, comme l'a dit très très bien Madame Préville c'est un amendement qui permettrait aux acheteurs publics de contractualiser des marchés publics de fournitures long terme d'énergie verte alors que les marchés publics de de fourniture d'énergie pourrait constituer un un véritable levier stratégique pour la transition environnementale ni l'article 15 du projet de loi ni les dispositions de la commande publique en vigueur ne permet aux acheteurs, il est temps, soumis de contribuer au déploiement des énergies renouvelables en effet aujourd'hui le droit de la commande publique, ne leur permet pas de s'engager dans le temps, lorsqu'il s'agit de fournitures courantes contraints d'acheter de telles fournitures sur une durée moyenne de 4 ans par la nécessité d'une remise en concurrence périodiques ces acheteurs n'ont pas la possibilité de permettre aux opérateurs économiques d'amortir dans le temps une infrastructure coûteuse nécessaires à la fourniture ou d'exiger que leur énergie soit produite par une nouvelle installation de production d'énergie renouvelable pour y remédier les est donc proposé de permettre à l'acheteur public pour la contractualisation d'un marché de fourniture en énergie renouvelable, issue d'un nouvel actif ne bénéficiant pas d'un soutien public et c'est important d'aligner la durée de son marché à celles de l'amortissement de l'investissement demandé aux producteurs d'énergie renouvelable, cela permettrait à ce dernier d'investir dans une nouvelle installation, en réduisant les aléas supporter et ainsi de rassurer ses partenaires et en particulier ses financeurs, j'ai beaucoup parlé pour dire finalement quelque chose de très, très simple, ces investissements s'amortit sur un temps long alors adaptons notre droit et nos possibilités de contractualisation à ces temps long. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. Oui, madame la présente les 2 amendements à 722 et. 1211 identique ne peuvent pas être retenu pour 2 raisons : la première, c'est que la prise en compte par l'État et les collectivités territoriales et de la diversification de notre mix énergétique et la promotion des territoires à énergie positive est déjà prévu parmi les objectifs généraux dans notre politique énergétique figurant aux articles L. 101 L 102 du code de l'énergie,

enfin, sur le plan juridique, le dispositif serait peu sûr car les objectifs prise en compte par les acteurs publics seraient très nombreux le code de l'énergie, y consacrant cathartique souvent large et parfois hétérogènes à ce sujet, il ne comporterait aucun délai d'application, de sorte qu'il pourrait avoir un impact négatif sur les contrats de fourniture d'énergie en cours, donc c'est une demande de retrait ou un avis défavorable de ces 2 amendements. Merci madame la ministre. le le rapporteur a effectivement si nous partageons un nouvel objectif parce que les acheteurs publics doivent contribuer au déploiement des énergies renouvelables, nous avons dans les mesures de simplification, récemment votée dans la loi ASAP en l'occurrence l'allongement de la durée des avances en compte courant et la possibilité d'alléger les exigences au titre au titre de la loi Sapin II des travaux qui sont également en cours pour mobiliser plus fortement le parc immobilier de l'État, à cette fin, l'article L 228 4 actuel il permet effectivement déjà de favoriser déploiement de du renouvelable dans la commande publique à travers l'expression de performance environnementale qui permet de favoriser les matériaux d'énergies renouvelables, qui ont la meilleure empreinte environnementale et puis le dans la rédaction même hein, de l'alinéa 2 qui vise l'article L 100 tirer 1 du code de l'énergie qui est beaucoup plus large que le seul développement des énergies renouvelables, le lien avec la commande publique serait difficilement opérationnel, c'est donc une demande de retrait sinon avis défavorable. Merci madame très ville Monsieur 2010 vous retirer. Vous mettez au revoir.

vote contre Ils ne sont pas adoptées, l'amendement 1083 monsieur Dantec. Ah non, pardon, ça que là il y a les Inuits merci madame. Présidente, mes chers collègues, cet amendement vise à rapprocher le débat d'entrée en vigueur de l'obligation d'introduire une part de matériaux biosourcés dans la commande publique d'utilisation de matériaux biosourcés concourent à la réduction sensible des émissions de gaz à effet de serre et à la préservation des ressources naturelles, la commande publique joue un rôle moteur dans le secteur de la construction et se doit d'être exemplaire en la matière, alors que la filière est déjà structurés pourquoi un telle attentisme cet amendement propose donc de rapprocher cette entrée en vigueur à 2023 et de renforcer, à l'horizon 2028 l'ambition jusqu'à 50 % de matériaux biosourcés dans les constructions et rénovations dans lesquels intervient la commande publique, je vous remercie. Merci madame la sénatrice poncer Mongin, monsieur le rapporteur.

je peux vous assurer, j'ai passé, nous avons passé beaucoup de temps à auditionner et toutes les entreprises que nous avons rencontrés ont une nécessité d'adaptation tant sur le des matériaux que sur la formation du personnel en 1er lieu la date de 2023 et trop rapprochés alors qu'elle celle prévue dans l'aérogare 1 sur ce sujet est fixé à 2030, on l'a évoqué tout à l'heure et en ce qu'ont lieu le pourcentage de 50 % est très élevé, tandis que la proportion envisagée par l'art va avoir sur ce point et plutôt de l'Ordre d'un quart à un tiers, donc cette demande de retrait ou un avis défavorable. Merci madame la ministre. je ne vous rejoins pas sur sa maturité, je pense qu'effectivement, comme vient de l'indiquer monsieur le rapporteur, cette filière, elle a besoin d'un temps d'adaptation qui est tout de même qu'il soit tout de même suffisant, malgré un fort volontarisme, on le sait, et donc sur cette période d'adaptation, je pense que l'horizon 2030 et et sincère et et raisonnables et que le calendrier que vous proposez à horizon 2023 serait trop contraint, c'est donc un avis défavorable. Merci madame la ministre, hein. Vous retirez je mais au je, mais voit donc la Mandement 846 avec 2 avis défavorables qui votent pour. pour. Abstention : il n'est pas adopté le 2 1093 Madame avait. Madame la présidente, cet amendement propose de revenir à l'esprit initial de l'article adopté à l'Assemblée nationale en focalisant l'obligation sur les matériaux biosourcés mais en ciblant sur les travaux de construction et rénovation lourde pour que cette obligation puisse prendre effet il est précisé que l'usage doit être significatif ce point il y a vocation à être précisées par décret, par ailleurs, l'amendement précise que l'obligation ne s'applique aux acheteurs publics au-dessus d'un certain seuil, à déterminer pour la cibler sur les acheteurs qui font régulièrement appel à des travaux de rénovation et de construction, je vous remercie. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. Oui, bien dans la présente. Le changement proposé par l'amendement n'est pas souhaitable d'une part il limiterait les matériaux promu à ce bio-sourcées faisant fi des matériaux Géo sur c'est au bas carbone, ce qui créerait une distorsion de concurrence que nous souhaitons pas d'autre part été établirait une référence aux rénovations lourdes, ce qui convient contreviendrait à la réglementation environnementale et romarin centrée sur les constructions, donc c'est une demande de retrait ou un avis défavorable. Merci madame la ministre. Cet amendement, il vise à revenir à la rédaction initiale qui a été votée par l'Assemblée nationale et qui étend la la rédaction de l'article L 228 4 du code de l'environnement, avec des objectifs, je crois, volontariste et ambitieux, les domaines d'application de cette mesure, ils concerneront la construction neuve, pour laquelle les exigences de la et revend auront déjà les faits recherchés mais aussi la rénovation lourde qui constituent un marché économique important pour les filières concernées, c'est donc par cet amendement qui prévoit d'encadrer par décret la mise en application de cette mesure, en particulier sur les seuils et la nature des travaux concernés, un avis favorable. Merci monsieur Dantec pour explication de vote. Oui, je pense qu'effectivement la la rédaction initiale et plus ambitieuse, donc nous allons évidemment la l'objectif étant qu'à la fin, nous ayons une CMP conclusive vont pas on prend que le mieux disant des 2 chambres, qui nous permettra de gagner quelques points, j'avais une question quand même un monsieur le rapporteur. La rénovation c'est beaucoup de l'isolation et les matériaux biosourcés sont particulièrement adaptés à la rénovation, donc je n'ai pas bien compris pourquoi écarter la rénovation alors qu'au contraire, en termes d'opportunité, il me semble que ça va de soi que c'est un des grands secteurs sur lesquels on a la possibilité, structurer rapidement une filière. Merci, je mets donc aux voix l'amendement 2000 93 avec un avis défavorable de la commission favorable du gouvernement qui vote pour. Qui vote contre.

au nom de la commission des affaires économiques le 1832. Oui mais a impression que j'ai très très rapide, qui est un amendement Rédac précision rédactionnelle. Merci madame la ministre. Pardon, je n'ai pas entendu, c'est un avis favorable, favorable. je mais voit cet amendement de précision qui vote pour. Contre, abstention il est adopté, je mets donc aux voix, l'article 15 ter ainsi modifiées qui votent pour contre. Abstention Abstention : il est adopté, nous passons à des articles additionnels le 467 monsieur Dantec. pour participer à la structuration de filière d'appliquer un taux réduit de TVA aux travaux d'entretien d'amélioration de réhabilitation de logements lorsque ceux-ci participent à la nécessaire transition écologique en utilisant des matériaux biosourcés ou le bois, il faut noter que tels taux réduit, a déjà été en vigueur de 99 à 2012, il avait été impressionné apprécié tant par les professionnels de la construction que par les particuliers, on comprend bien qu'effectivement ça réduit le coût pour les particuliers et pour tous les particuliers, quelle que soit leur revenu, à la différence du système qui existe dans un ma prime, alors j'ai bien entendu un monsieur le rapporteur, ça nous permettra peut-être de répondre à ma question précédente en même temps, disant que c'était trop tôt pour les professionnels, d'avoir une filière complète, mais rien n'empêche quand même d'aider à ce qu'elle structure le plus vite possible et créer un appel, un appel d'air par les travaux, donc je crois que c'est assez cohérent avec l'endroit où nous voulons arriver en 2003. Merci, cher collègue, l'amendement 189 madame. Merci madame la présidente, nous le savons, le secteur du bâtiment et le 2ème secteur émetteur de gaz à effet de serre en France au-delà des des actions qui doivent être engagées pour concourir à la réduction des consommations énergétiques des bâtiments, une attention particulière doit être portée aux techniques constructives, bien évidemment, et plus particulièrement aux matériaux utilisés, en effet, on le sait, le béton est produit à partir de ciment, dont la production représente à elle seule de 5 à 7 % des émissions globales de gaz à effet de serre dans le monde, les actions doivent être donc conduite conduite afin d'inciter à l'utilisation des matériaux biosourcés des mesures doivent être prises, touchant l'ensemble des bâtiments logements privés et publics, bâtiments publics et privés à usage professionnel, c'est pourquoi, dans un souci de lisibilité de simplification, nous proposons d'abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable à l'acquisition de matériaux biosourcés cet amendement, nous le déposons régulièrement son adoption pourrait trouver toute sa place dans ce projet de loi de transition écologique. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. Oui, madame la présidente, madame ami sur collègue ces 2 amendements en objet similaire il lui vise à réduire le taux de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est une idée intéressante, mais cette proposition n'est pas opportune pour 3 raisons : la première, c'est que la réduction de taux de TVA sont strictement encadrées par le droit, l'Union européenne, la 2ème, c'est qu'il existe déjà des taux réduit de 5 5 à 10 % sur les opérations de rénovation énergétique ou de construction et la 3ème, en ciblant les matériaux bio-sourcées à l'exclusion de ce ressourcer ou bas carbone le dispositif introduirait une distorsion de concurrence entre les différentes filières, des matériaux de construction, j'en profite pour répondre en même temps, avant notre collègue Dantec où j'allais pas pendu tout à l'heure, nous voulons pas instaurer de distorsion de concurrence à travers ses différents matériaux, donc c'est une demande de retrait sinon avis défavorable.

de la taxe sur la valeur ajoutée, donc contraire au au droit de l'Union européenne et puis d'une manière générale, je, je renverrai aisément ce ce débat fiscal à nos travaux sur le projet de loi de finances merci défavorable.

Abstention : il n'est pas adopté même vote pour le 189 votes, il ne doit pas adoptée nous fait son à l'amendement 466 présenté par Monsieur Dantec. j'espère que nous tous nos taux réduit de TVA à 5 5 ne vont pas passer à la trappe parce qu'on en a voté un de manière assez consensuelle concernant le rail et le le ferroviaire, c'est quand même un outil que nous ne détestons pas utiliser et dans les propositions pour l'utiliser parce qu'on sait que c'est quand même un outil très puissant, nous vous proposons donc de l'utiliser pour ce qui est de l'utilisation de bois en provenance de forêts exploitées durablement et de favoriser ainsi la relance économique, de la foresterie local et national, donc c'est une proposition qui va dans le sens, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en discuter après d'utiliser au mieux les ressources de la forêt française enlacés sous et mal exploité : on sait qu'on a là un enjeu majeur qu'on a un enjeu majeur aussi de sécurisation aujourd'hui de notre production de bois beaucoup d'artisans, la presse en effet beaucoup écho se plaignent aujourd'hui de la de la pénurie sur le le bois, donc, dans, dans le cas de sa structuration meilleur de l'exploitation de la forêt française qui est une opportunité de stockage de de carbone à travers la construction bois un notamment ce taux de TVA à 5 5 serait tout à fait opportun. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. Oui, madame la présidente, hélas, mon cher collègue, on est dans la même situation du droit, l'Union européenne sur la TVA, puis la 2ème raison qui pose un autre un autre souci, c'est que vous faites un une séparation en fonction des espèces des variétés de bois qui pourraient en bénéficier et et là il y a un risque vraiment important d'inconstitutionnalité au niveau de 1 tels amendements, donc c'est un avis et demande de retrait ou avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Effectivement, nuance sur sur le bois de chauffage en dehors de ce bois de chauffage, le droit européen qui régit la TVA n'autorise pas l'application de 2 taux réduits au bois, donc c'est un un avis à nouveau défavorable. remercie, je mets donc on voit cet amendement avec 2 avis défavorables qui vote pour. Contre, abstention, il n'est pas adopté, nous passons à la discussion commune de cet amendement le 1976 monsieur Cabanel. madame la messe madame la Ministre et cher collègue, les grandes entreprises françaises doivent prendre leur part dans la transition écologique et adapter leur modèle d'affaires afin de le rendre plus résiliente face au dérèglement climatique, le président Herman demain vise à rendre obligatoire la publication annuelle par les grandes entreprises de rapport Climat annexé la déclaration de performance extra-financière ce rapport Climat permettrait aux sociétés concernées de présenter leur engagement en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de C1 compatible avec la stratégie bas carbone et l'accord de Paris les engagements seraient pris sur la base d'un bilan démission complet d'une trajectoire de réduction standardisé et d'un plan d'investissement compatibles.

Merci madame la présidente, afin de respecter nos engagements climatiques, les grandes entreprises françaises doivent prendre toute leur part dans la transition écologique et adapter leur modèle d'affaires pour être plus résiliant au regard des enjeux environnementaux pour permettent d'anticiper les différents impacts du dérèglement climatique, cet amendement tend favoriser la transparence sur la transition des grandes entreprises vers une économie bas carbone renforcer la qualité et la comparabilité de la donner extra-financière permet d'améliorer la robustesse de robustesse de l'ensemble des analyses qui en découlent et donc de mieux orienter les flux financiers comme de crédibiliser les engagements pris par les acteurs financiers sur le plan réglementaire, la France a été à l'avant-garde sur le sujet de la publication extra-financière des entreprises et des investisseurs, avec l'article 116 de la loi nouvelles régulations économiques promulguées dès 2001, nous devons capitaliser maintenir cette avance et nous positionner en Europe et dans le monde, savoir mesurer les impacts environnementaux devient aujourd'hui une compétence critique en amont de la révision de la directive sur le reporting des données extra-financière, la France doit être exemplaire en matière de transparence de ces données, cet amendement prévoit donc que les sociétés soumises à l'obligation de déclaration de performance extra-financière soit soumise à l'obligation de publication d'un rapport Climat : je vous remercie. Merci, cher collègue, l'amendement. Numéro 1768 qui n'est pas défendu l'amendement 1975 monsieur Cabanel. C'est un amendement identique donc défendu merci. merci. Si cher collègue, l'amendement 808 Monsieur Gay. Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cet amendement transcrit dans notre droit, 2 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, il a pour objet d'inclure les émissions indirectes au bilan d'émissions de gaz à effet de serre, dit de Scop 2 et 3, soit celles issues de la consommation énergétique ou l'utilisation des produits énergie de rendre obligatoire la tenue d'un hôtel bilan pour toutes les entreprises, celles de moins de 500 salariés seraient cantonnés à des obligations plus légère, 3 de conditionner les aides publiques au respect de la trajectoire fixée par ces entreprises, et enfin pour finir, nous proposons que les sanctions ne seront plus plafonnées à 10000 euros mais à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos je vous remercie. Si cher collègue, enfin, l'amendement 1511 présenté par Madame Bricq. Merci madame la présidente, notre amendement propose de conditionner l'ensemble des aides publiques perçues par les entreprises au respect d'un socle minimal en matière de respect de l'environnement de transparence fiscale et de devoir de vigilance les entreprises seraient concernées en fonction d'un chiffre d'affaires dans le seuil serait fixé par décret, très concrètement, cet amendement impose aux sociétés bénéficiaires d'aides publiques, de respecter les dispositions de l'accord de Paris sur le climat et de remettre chaque année un rapport sur la trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, il prévoit également que ces mêmes sociétés ne détiennent pas d'actifs dans les paradis fiscaux et qu'elles respectent leur devoir de vigilance, la solidarité nationale est ainsi conditionnées à une responsabilité environnementale, sociale, mais aussi fiscales des sociétés bénéficiaires des aides publiques, l'adoption de cet amendement serait un gage forts traduisant réellement la volonté de verdissement de notre économie affichés dans ce projet de loi, je vous remercie. Merci, cher collègue, monsieur le rapporteur, votre avis sur ces différents amendements. S'il vous plaît, merci madame la présidente, non plus les cet amendement si j'ai bien noté mais les 5 amendements, c'est bien cela. Alors l'article L 225 tiré sans de tirer un du Code du commerce dispose déjà que la déclaration des performance extra-financière des entreprises, je cite, comprend notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, l'annexion d'un rapport Climat présentant la trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, assortie d'une amende en cas de non-publication et source potentiellement de charges nouvelles pour les entreprises. Plutôt qu'une démarche vertical, il est préférable de mettre en oeuvre un système incitatif qui responsabilise les entreprises si sur le fond, a-t-elle rapport présente une utilité certaine la manière dont cette obligation nouvelle s'intègre dans notre droit n'est pas satisfaisante, il est donc proposé un avis défavorable sur l'amendement 1976 et les amendements identiques 776 et 1975 avis défavorable également sur les amendements 808 et 1511 prévoyant une conditionnalité environnementale dans le versement des aides publiques. Merci, monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. le, sur l'amendement les amendements qui visent à compléter la déclaration de performance extra- financière en introduisant la publication d'un d'un rapport Climat annuel une une trajectoire qui serait fixé de réduction des gaz à effet de serre, avec un suivi dans le temps, en cohérence avec la SNPC et l'accord de Paris je crois que faire progresser la prise en considération des enjeux climatiques et la transparence sur ces mesures, bien sûr, évidemment nous partageons ce ce souci avec un droit en vigueur, d'ailleurs, qui répond déjà en partie à ces préoccupations, puisqu'un bilan des émissions de gaz à effet de serre est prévue à l'article L 229 25 du code de l'environnement, il doit être publié chaque année par les entreprises de plus de 500 salariés et être accompagnée d'un plan de transition qui présente les objectifs, les moyens et les actions envisagées et puis le cas échéant les actions évidemment mise en oeuvre, l'article 244 de la loi de finances initiale pour 2021, il prévoit, lui, d'appliquer un dispositif similaire mais simplifiée pour les entreprises de plus de 50 salariés qui seraient bénéficiaires d'aide directe au titre du plan de relance donc le dispositif qui est qui est proposé un largement apparaît comme excessivement complexe et difficile à à mettre en oeuvre, notamment dans la dans ce qui concerne les contrôles et les sanctions avec d'ailleurs un cadre réglementaire de la DPE est ce qui est déjà très complexe et en cours d'évolution au niveau européen, donc dans le cadre des travaux préparatoires de la révision de la directive sur le reporting extra- financier cette possibilité d'inclure les obligations de reporting liés à la prise en compte par les entreprises de l'accord de Paris est envisagée et ce sujet de la planification de la réduction des émissions, il pourra donc plus efficacement être approfondie dans le cadre de ces négociations européennes, je vous propose donc de ne pas préempter c'est ces dispositions au niveau national, ce sera donc sur ces amendements, un avis défavorable, comme sur le 15 11 de la sénatrice briquet sur ce ce cet amendement qui vise à conditionner le versement d'aides publiques à la définition annuel de de trajectoire de réduction des émissions qui présente un certain nombre de difficultés pratiques, hein, d'une part dans la notion de respect des dispositions de l'accord de Paris qui n'est pas définie à la main et de l'entreprise et donc là où il n'existe pas de méthode reconnue pour décliner ses ses engagements à l'échelle de l'entreprise et puis par ailleurs avec une mesure que vous proposez, qui s'appliquerait, quel que soit le type de subventions versées donc quel que soit son montant, y compris donc pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire, ce qui semble évidemment et excessif dans le contexte sur le l'amendement 808 concernant la généralisation et de la prise en compte de l'ensemble des émissions directes et indirectes, et donc des émissions indirectes non associés à l'énergie dite du scope 3 il est rappelé que cette disposition avait déjà porté par le projet de décret qui est relatif au bilan d'émissions de gaz à effet de serre dont la consultation du public par internet s'est déroulé du 19 le Conseil d'État sur la réalisation d'un bilan d'émissions simplifié qui portera uniquement sur les émissions en Direct des personnes morales de droit privé de moins de 500 salariés, l'article 244 de la loi de finances pour 2021, qui instaure la réalisation d'un bilan simplifié pour les entreprises de plus de 50 salariés répond en partie aux demandes concernant l'extension des 10. Positif aux plus petites entreprises, enfin sur la conditionnalité du versement d'aides publiques aux résultats du bilan d'émissions, la fixation de critères systématique, elle serait complexe, elle est très sensible, où vous le savez, dans le contexte de relance économique, les conditions de versement des aides publiques, elles sont propres à chaque dispositif, ce qui permet de tenir compte de la diversité des aides publiques existantes, je crois que nous devons garder cette cette nuance et surtout. Cette cette réactivité, réactivité, cette souplesse dans le contexte de crise économique que nous savons, c'est donc un avis également défavorable. Un avis défavorable pour tous les amendements, que ce soit de la commission ou du gouvernement, donc nous allons mettre voix ces différents amendements avec 2 avis défavorables. Commission et le gouvernement pour chacun le 1976. Je mets aux voix qui vote pour. Contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté 2 identiques 776975 2 avis défavorables qui vote pour. Contre qui s'abstient, ils ne sont pas adoptés le 808 même combat, il n'est pas adopté le MD 11 même vote pas adopté.

Que la déclaration de performance extra-financière des entreprises présentes concrètement l'apport de leurs activités à l'atteinte des engagements pris par la France en faveur du climat et notamment les objectifs de développement de développement durable, telle qu'adoptée par l'Assemblée générale des Nations-Unies, le 25 septembre 2015, les objectifs de développement durable, pourrait ainsi devenir une grille de référence commune pour l'ensemble des entreprises et contribuer à faire progresser les politiques RSE, cela nous semble nécessaire au regard des transformations profondes qu'elles doivent engager, nous proposons à titre à ce titre d'introduire dans ce projet de loi un chapitre dédié au renforcement de l'engagement environnemental des entreprises, je voudrais faire une petite parenthèse, parce que c'est vrai que les objectifs du développement durable s'impose de plus en plus dans le dans le débat parlementaire et nos collègues de l'Assemblée nationale ont d'ailleurs adopté en décembre dernier une résolution pour intégrer ces objectifs dans la Constitution. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente, alors sans reprend des arguments, j'ai pu développer il y a quelques minutes sur les amendements votés à l'instant, en faisant référence toujours au même article, à savoir la. L 225 tirer un du Code du commerce vous dire simplement que cette obligation d'intégration des objectifs de développement durable à la déclaration de performance extra-financière des entreprises n'ajoute rien de substantiel par rapport au droit existant et présente surtout une portée déclaratoire les entreprises sont actuellement de se référer ou non aux objectifs de développement durable à rendre obligatoire, soit une source de complexité supplémentaire qui n'est pas au opportun d'introduire et donc c'est un avis défavorable qui est proposé. Merci, Madame le Ministre.

plus nous en sortirons grandis et renforcés, c'est d'ailleurs effectivement, vous l'avez dit, ce que l'Assemblée nationale a fait en adoptant une une motion il y a quelques mois maintenant, nous l'avons fait et vous l'avez fait avec l'article 15 qui sur la commande publique intègre plusieurs mentions et références aux aux nous l'inscrivons donc dans le dur, si j'ose dire et et dans le droit, et c'est tant mieux ici, donc vous savez la déclaration de performance extra-financière, elle est réglementée au niveau européen, actuellement des travaux de révision de la directive de 2014 ont lieu sont en cours et un projet de directive donc c'est SRD d'avril 2021 va nous amener à intégrer, et vous le savez, la France est moteur dans ces négociations, ces ces critères et ses références dans les négociations européennes, c'est donc une demande de retrait à défaut : avis défavorable. Merci madame la ministre, je vais donc on voit cet amendement avec 2 avis défavorables à qui vote pour. pour. Abstention : il n'est pas adopté, nous passons maintenant à une discussion de trois amendements d'une discussion commune, nous avons d'abord 2 amendements identiques : le 870 madame ses manches. Merci madame la présidente, cet amendement vise à faire évoluer la déclaration de performance extra-financière vers une déclaration de performance intégrées en rendant obligatoire la publication par les entreprises, des informations sur les moyens financiers qu'elle mobilise pour la préservation de l'environnement, comme le demandait la Convention citoyenne pour le climat lorsque souhaitait renforcer les obligations relatives aux exigences environnementales des entreprises, les réglementations européenne et française oblige, les grandes entreprises à publier un certain nombre d'informations concernant les politiques environnementales et sociales le problème en en l'état, c'est que les informations environnementales sont décorrélées des informations financières et ne permettent ainsi ni d'estimer l'engagement réel des sociétés au regard des politiques en matière d'environnement ni de mettre en place des mécanismes incitatifs efficace notamment fiscaux en faveur de la transition écologique donc une telle évolution de la déclaration de performance extra-financière vers la déclaration de performance intégrées doit permettre à la fois de faire la transparence sur les coûts environnementaux engagés par les entreprises sur leur exercice passé et de fournir des informations sur les coûts environnementaux budgétés pour les exercer si à venir et donc de lire l'évolution des politiques de l'entreprise en matière d'investissement cette évolution vers une des pays traduira les responsabilités des entreprises vis-à-vis de la crise écologique, ces coûts environnementaux devront recouvrir à la fois les dépenses environnementales, soit les dépenses mobilisés par l'entreprise pour prévenir, réduire ou réparer les dommages qu'elle cause à l'environnement mais aussi les dépenses en faveur de la transition écologique qui soit : les dépenses visant à réorienter écologiquement son modèle d'affaires ces propositions s'appuie en grande partie sur des recommandations du Conseil national de la compacte, comptabilité et de l'Autorité des marchés financiers, paru en 2020 en 2003, elles n'ont pourtant jamais ou très peu étaient mises en pratique, alors que cette mesure devrait faire consensus dans le cas de la transition écologique, je vous remercie.

a été, il a été défendu, hein, c'est le même amendement qui vise à faire évoluer la déclaration de performance extra-financière vers une déclaration de performance intégrées. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis sur ces trois amendements. Merci madame la présidente, donc c'est ce sera un avis défavorable pour les mêmes raisons que j'ai pu développer il y a quelques minutes sur les aime les amendements précédents.

les travaux de révision qu'on a évoqué et la directive s'est SRD doit permettre ces ajustements et dans le même temps, nous devons approfondir dans le cadre de ces négociations, les échanges, le débat le partage sur ces nouvelles dispositions avec les parties concernées, je pense en 1er lieu aux professions comptables aux fédérations professionnelles, en l'état, parce que la perspective est très intéressante : une demande de retrait sinon avis défavorable. Merci, je mets donc aux voix les 2 amendements identiques 870977 avec 2 avis défavorables qui vote pour.

Merci madame la présidente, chaque projet de loi de finances vient ajouter de nouvelles strates d'aides publiques aux entreprises, au point qu'elle qui elles-mêmes font régulièrement appel à des cabinets d'expertise, spécialisé dans l'optimisation d'aides publiques ce brouillard et non seulement source d'inégalité entre les grandes entreprises qui ont les moyens et le temps de réaliser les démarches mais il est surtout dommageable car il constitue pour de nombreux crédits d'impôts et d'aides, peu ou pas conditionnée à des comportements vertueux un levier manque manquer pour la transition écologique, cet amendement reprend la première propositions du rapport d'information de l'Assemblée nationale sur la conditionnalité des aides publiques, il vise à instituer au sein du Parlement un office parlementaire commun d'évaluation des aides publiques nationales aux entreprises, ce dernier serait chargée de l'évaluation et du suivi des aides publiques et de leur conditionnalité, parmi lesquels les comptes dossier conditionnalité environnementale, ils seraient habilités à adresser à la Cour des comptes, une demande d'enquête ou d'évaluation sur des aides publiques spécifique réservée à ce jour à la commission des finances à la commission des affaires sociales aux commissions d'enquête et aux présidents des assemblées cette faculté de saisine permettrait à l'Office de bénéficier d'un éclairage et d'une assistance dans ses travaux d'évaluation. Merci à vous. L'idée d'un office parlementaire d'évaluation des aides publiques nationales aux entreprises est intéressante, cependant, cependant elle repose sur la création d'un nouvel organe parlementaire commun aux 2 assemblées, alors que le Sénat dispose déjà d'une délégation d'entreprises qui pourrait être confié ces missions sans qu'il soit besoin de créer une nouvelle instance ad-hoc en conséquence c'est un avis défavorable qui est proposé. Merci madame la Ministre. Mais sur le fond, je rejoins monsieur le rapporteur sur la forme, effectivement, on peut considérer que ce sont aux chambres de se prononcer sur leur propre organisation je rejoindrais donc l'avis défavorable.

Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, donc le le rapport de la Convention citoyenne pour le climat qui a été donc adopté le 21 juin 2020, a rappelé que la transition écologique ne peut constituer une opportunité pour l'économie et l'emploi, que si des dispositifs d'accompagnement adaptés sont mis en oeuvre à destination des salariés et des entreprises, la Convention citoyenne pour le climat a également fixé comme l'un de ses objectifs phares: l'accompagnement à la reconversion des entreprises et des salariés pour faire évoluer leurs activités, voire en danger si elle devait disparaître certains secteurs d'activités comme le secteur automobile ou le secteur aérien sont aujourd'hui contraints de repenser en profondeur leur modèle économique pour répondre à l'urgence écologique, les conséquences économiques et sociales de ce basculement vers un nouveau modèle économique décarbonés doivent donc être anticipé notre amendement demande au gouvernement de mettre en oeuvre une stratégie nationale concertée de programmation des emplois et des compétences de la transition écologique pour la période 2022 2023, cette stratégie est nécessaire pour identifier et accompagner l'évolution des métiers et des compétences et des formations de la transition énergétique pour définir les priorités d'action pour anticiper les besoins des entreprises et pour mettre en place les reconversions professionnelles qui sont induites cette stratégie doit être concertée opérationnel, elle doit aborder concrètement les besoins en financement définir le pilotage des actions à mener pour certaines de plus au plus près des territoires et proposer des indicateurs et des outils de suivi partagé cette stratégie serait le pendant, employes de notre stratégie bas carbone, enfin, cette mesure permettrait de donner des perspectives en matière d'emploi et de la consistance à un projet de loi qui affiche l'ambition d'adapter l'emploi à la transition écologique et nous ne partons pas de rien, puisque le doigt citer le plan de programmation des emplois et des compétences, pour lequel une mission de préparation avait été confiée à Madame Laurence Parisot et ce rapport déjà été rendu il y a maintenant plus de 2 ans parce qu'il était rendu le 19 février 2019, donc nous avons tous les éléments pour que cette stratégie concertée puisse être mise en oeuvre. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. Même si nous pouvons partager l'objectif de cet amendement ce ce dernier consistant à créer une stratégie nationale concertée de programmation des emplois et des compétences de la transition écologique me semble constituer une injonction formulée à l'égard du gouvernement, ce qui n'est pas conforme à notre constitution, et donc c'est un avis défavorable qui est proposé. Merci madame la ministre. Merci de d'avoir cette à cette attention par ailleurs je pense que de nombreux outils hein, qui sont portées par le ministère de la transition écologique, le ministère du Travail Laden l'Observatoire national de l'emploi et des métiers de l'économie verte ou encore France Stratégie ils permettent de réaliser ces travaux d'anticipation et d'accompagnement des des entreprises et des salariés dans la transition avec d'ailleurs des dispositions qui sont prises dans ce projet de loi climat résilience qui va permette de renforcer la prise en compte de la transition dans les négociations collectives avec les partenaires sociaux qui pourront, dans ce cadre, se concerter pour anticiper les évolutions et mettre en place et les formations adéquates, donc nous avons ici avec des opérateurs qui pourront accompagner les branches et les entreprises dans ses démarches, des outils qui sont déjà, je crois, largement mobilisables, c'est donc un avis défavorable. Merci monsieur Dantec avec pour explication de vote. Oui, donc je viens d'entendre Madame la Ministre, France Stratégie c'est une bonne idée, donc où est le rapport de France Stratégie qui nous permet d'analyser le projet de loi de climat qui est aujourd'hui au Parlement. la logique aurait été que cette mobilisation elle aient lieu en amont de la discussion du projet de loi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on a aussi un nouveau commissariat au Plan, vous n'avez pas mis dans l'énumération

on a maintenant un objectif quantitatif mais où on veut aller sur l'industrie automobile sur les industries des énergies renouvelables, on a voté collectivement tout à l'heure un amendement intéressant sur une stratégie d'entreprise photovoltaïque, mais tout ça, c'est totalement épars, on a des éléments d'un puzzle on n'a pas de vision globale, on n'a pas de vision globale non plus sur les outils financiers, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure par rapport à la Caisse des dépôts, il est quand même temps qu'on ait cette stratégie, donc je pense que cet amendement et questionne, il essaye de répondre à ça, nous n'avons pas de véritables stratégies aujourd'hui et c'est pour ça que nous ne pourrons pas tenir nos engagements climat en l'état actuel des choses. Merci monsieur le pour explication de vote. Merci madame la présidente, je voudrais vous avez Madame la Ministre, que je ne comprends pas votre réponse, c'est-à-dire qu'on on confie il y a 2 ans, un rapport à Madame Parisot qui on peut pas reprocher forme d'impartialité politique, bien au contraire, je crois que la lucidité du rapport, c'est bien de définir quels sont les secteurs d'activités qui vont évoluer, de les quantifier, de faire ce qu'il faut ce qu'il faut faire de faire d'un certain nombre de recommandations, il y a, il y a une douzaine de recommandations et puis ce rapport hé bien visiblement, il reste dans les cartons, il ne débouche pas sur ce qu'il devrait déboucher, c'est-à-dire une cohérence par rapport à cette programmation des emplois et des compétences qui vont être lourdement impacté par la transition écologique. Merci, je mets donc on voit cet amendement 1513 avec 2 avis défavorables qui vote pour.

L'atteinte de nos objectifs climatiques implique une transformation profonde et inédite de nos manières de nous déplacer de produire, de nous loger de nous nourrir, en fait, il faut avoir une vision, comme vient de le dire Monsieur notre économie va nécessiter le déploiement d'emplois dits verts, c'est-à-dire compatibles avec la transition écologique parmi ces emplois verts Les Échos en activité qui produisent des biens ou services ayant pour finalité la protection de l'environnement ou la gestion des ressources qui mobilise aujourd'hui 1,8 % de l'emploi en France, elle concerne l'agriculture biologique, la protection de la nature des paysages et de la biodiversité, le recyclage, la récupération des eaux, la recherche et le développement encore l'ingénierie des énergies renouvelables, de nouvelles compétences vont donc se déployer dans les prochaines années, mais déjà un certain nombre d'emplois peuvent être rapidement créée localement en fonction des besoins identifiés dans chaque bassin de vie, ces emplois peuvent être portés par des entreprises, des administrations ou des structures de l'économie sociale et solidaire, un 1000000 d'emplois pourraient être créés pour un coût inférieur aux politiques de lutte contre le chômage existantes, à l'heure actuelle, nous pensons que l'État et les collectivités doivent s'engager dans une démarche innovante permettant d'adapter réellement l'emploi à la transition écologique cette question mérite davantage qu'un simple affichage dans un projet de loi pour embarquer tous les citoyens dans la dynamique de transition écologique et faciliter son acceptation sociale, l'état de pouvoir offrir aux Français des perspectives et opportunités nouvelles, notamment en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi aujourd'hui, nous considérons que cette approche inclusive et solidaire est le préalable à toute transition écologique d'envergure, le délai d'essayer au gouvernement pour présenter ce rapport est volontairement court, car d'une part des propositions sont déjà sur la table et d'autre part, il convient d'être prêt pour proposer des ajustements nécessaires lors des prochaines lois de finances nous considérons en effet qu'il y a urgence à mobiliser les citoyens et les acteurs de terrain autour de ce projet porteur pour notre pays, je vous remercie. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur, votre avis. Merci madame la présidente, ce d'amendement propose la remise au Parlement d'un rapport proposant les mécanismes de création de financement et de déploiement d'un dispositif de garantie à l'emploi Vert, je ne suis pas favorable à multiplier les demandes de rapport demande déjà très nombreuses dans ce projet de loi et c'est donc un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, Madame le Ministre. Je rejoindrais le souci de monsieur le rapporteur, même si, effectivement, nous avons déjà un des travaux sur ce sur ce thème et surtout un dispositif territoires zéro, chômeur de longue durée que la loi du 14 décembre dernier qui a été votée à l'unanimité au Parlement. Prolongée qui a prévu d'éteindre le dispositif avec un élargissement, vous le savez des 10 territoires actuellement expérimenté à 50 nouveaux territoires et qui est très largement inspiré de ce dispositif, donc un retour sur expérience qui nous permet largement d'éclairer votre. Votre demande avec de nombreux emplois qui sont créés dans ce cadre, je vous propose donc que nous suivions l'extension de cette expérimentation avec la plus grande attention et que nous nous basons sur ses réflexions, c'était un avis défavorable. Merci madame la ministre, je mets donc aux voix cet amendement il 514 avec 2 avis défavorables qui vote pour.

Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes avec cet article 16 au coeur du titre produire et et travailler ce type n'est pas neutre parce que l'industrie représente 17 % des émissions de gaz à effet de serre et qu'elle doit réduire ses émissions de 81 % en 2050 selon la stratégie nationale bas carbone, cela suppose que nous devons produire et travailler différemment pour surmonter ce défi qui ne sera pas et on l'a déjà vu sans conséquence sur l'emploi et et sur les compétences, d'où la nécessité, comme on l'a dit tout à l'heure de prévoir d'anticiper et d'accompagner cela avec une stratégie nationale mais aussi, et, et, là aussi, nous en avons encore parler d'un volontarisme pour satisfaire les besoins vers les nouveaux emplois verts de la transition écologique mais la réussite des objectifs se fera avec le concours de tous, des chefs d'entreprise mais aussi bien évidemment des salariés plusieurs leviers peuvent être mobilisés le statut d'entreprise à mission afin de permettre à ces dernières de s'inscrire dans des stratégies gagnantes sur le long terme avec des finalités d'ordre social ou environnemental pour préserver ses entreprises de l'opportunisme vorace de certains fonds de pension qui recherchent malheureusement la rentabilité à court terme 2ème levier, c'est la négociation collective, dans le cas de la gestion des emplois et des parcours professionnels, enfin le 3ème c'est avec le comité social et économique de l'entreprise qui doit se voir attribuer des compétences pour traiter des conséquences environnementales des activités de l'entreprise et pour lequel les représentants des salariés doivent être dotées de moyens complémentaires, y compris en formation pour appréhender ces sujets, faisons confiance au dialogue social à la négociation à l'implication des salariés pour mieux accompagner nos entreprises à relever les défis de la transition écologique et ce sera le sens des amendements que nous avons déposé et que nous aurons à coeur d'examiner tout à l'heure. Merci, cher collègue, la parole est à présent aux sénatoriales. Merci madame la présidente, madame la Ministre, mes chers collègues. La crise sanitaire va, malheureusement, conduire à la suppression de dizaines voire de centaines de milliers d'emplois, il apparaît donc urgent de mieux répartir le temps de travail en réduisant le temps hebdomadaire travaillées par toutes et tous, mieux et moins travailler pour mieux et travailler toutes et tous la Convention citoyenne pour le climat avait d'ailleurs dans un 1er temps retenu cette proposition de réduire le temps de travail à 28 heures hebdomadaires pour notre part, nous proposons seulement 32 heures mais avec une campagne médiatique extrêmement forte d'une partie du patronat et du gouvernement, opposé à la réduction du temps de travail, la convention climat a reculé sur cette mesure, nous regrettons pour notre part que nos amendements proposant la baisse du temps de travail et étaient considérés comme des cavaliers législatifs, qu'une étude récente, publiée par le Guardian a rappelé l'impact de notre temps de travail sur le dérèglement climatique, selon cette étude, nos temps de travail influence largement le réchauffement climatique, et cela s'explique par les déplacements en voiture, mais également par la production de biens de consommation et par l'envoi de mails en bref moins travailler permettrait de réduire notre utilisation de ressources, la durabilité écologique nécessite une baisse générale de la consommation et l'augmentation du temps de loisirs n'est pas un luxe mais une urgence grâce aux progrès technologiques et à l'augmentation de la productivité, nous pouvons nous interroger sur l'utilisation du temps gagné, nous posons la question du partage de la productivité et de l'amélioration de la qualité de vie des salariés, la baisse du nombre d'heures de travail par semaine tout en maintenant les rémunérations permettrait d'agir sur les conditions de travail, l'épanouissement personnel, favoriser l'embauche et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis ce que je vois qu'il y a beaucoup de brouillard et que vous avez donc beaucoup d'arguments à m'opposer à cette question du tram travail moi je regrette une chose pourquoi vous ne l'avez pas accepter les amendements et puis après, il y aurait eu un vote, mais surtout un débat parce que je vois qu'il y a beaucoup d'arguments, je les entends là mais j'aurais préféré les entendre au micro : je vous remercie. Merci, chers collègues, nous abordons l'amendement numéro 21 52 présenté par le gouvernement, Madame le Ministre. Merci madame la présidente, en rétablissant les dispositions qui prévoient la prise en compte des enjeux de transition écologique dans les dispositions supplétives relatives à la négociation concernant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, tant au niveau de la branche que des entreprises d'au moins 300 salariés est proposé, qui a été proposé en commission au Sénat, elle remet en question l'esprit des ordonnances de 2017 qui consiste vraiment à circonscrire les dispositions d'ordre public aux obligations et thématique générale de la négociation collective en entreprise lorsqu'il s'agit de préciser un thème de négociation ou d'ajouter un sous-thèmes il rajouter systématiquement dans les dispositions supplétives afin d'une part, de ne pas alourdir les obligations d'ordre. Public et, d'autre part de renforcer l'incitation des partenaires sociaux à conclure des accords de méthode qui organise la négociation collective, dans les faits en vue du très faible nombre d'accords de méthode conclu sur le fondement des dispositions d'ordre public, ce sont des dispositions supplétives qui trouveront sans doute principalement à s'appliquer et puis d'autre part, cet amendement il rétabli des dispositions concernant les attributions du comité social et économique avec une modification qui a été proposé en commission qui supprime toutes les dispositions de l'article 16 relative à la consultation du CSE sur les enjeux environnementaux et qui remet donc en cause le l'objet même hein et les dispositions du présent projet de loi, c'est pourquoi le gouvernement se propose le rétablissement de ces dispositions pour enclencher une dynamique vertueuse, je crois que c'est une les enjeux environnementaux, c'est une préoccupation qui est largement partagée au sein de l'entreprise, c'est un objet de dialogue social, ces dispositions à 5 rive, elles s'inscrivent en parfaite cohérence avec les propositions de la Convention citoyenne qui souhaite l'adoption d'une mesure législative destinée à élargir les missions du CSE elle n'entraîne aucun coût simplement elles élargissent et elles intègrent ces réflexions, je vous demande donc si vous voulez bien de, de, d'accepter de rétablir ces dispositions. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ce cet amendement du gouvernement. Merci madame la présidente, cet amendement du gouvernement, a pour objet donc de rétablir, comme vous venez de le préciser, Madame la ministre, l'article dans sa version adoptée à l'Assemblée nationale, la commission notre commission a supprimé certaines dispositions de l'article 16 difficilement intelligible et qui confie au comité social et économique des missions qui ne relève pas de sa fonction, les comités sociaux économiques ont été mises en place suite à l'une des ordonnances du 22 septembre 2017 il semble prématuré d'élargir leur mission alors qu'ils peinent encore à se saisir de la plénitude de leurs attributions en outre les réformes récentes ont cherché à laisser davantage les acteurs de l'entreprise définir leur agenda social en levant des contraintes juridiques, conduisant à des consultations uniquement formelle cet article va à l'encontre de cette dynamique et donc, la commission propose d'émettre un avis défavorable. Je vous remercie, monsieur le rapporteur monsieur Dantec. nous nous voterons bien sûr pour pour rétablir non, l'ambition initiale du du du texte, il se trouve que je je discutais ce week- end avec le directeur d'une d'une très grande école française qui me disaient que, aujourd'hui, ces étudiants ont tendance à choisir plutôt des PME que les grandes entreprises habituel qui jusqu'à présent étaient plutôt la la voie royale pour beaucoup des d'étudiants de grandes écoles et il me disait derrière que c'était par rapport à une quête de sens, je pense que ce qui se joue dans notre discussion à ce niveau-là, c'est justement le sens du travail dans l'entreprise et le fait d'ouvrir les débats du comité social et économique effectivement à l'ensemble des impacts de l'entreprise et à sa part de la responsabilité globale, parce que tout ce qu'on fait depuis le début de ce texte d'assumer notre petite part à chacun de la responsabilité globale et d'organiser l'action collective à partir de là je je crois qu'effectivement donné au CSE, un rôle dans ce débat éclairé les salariés sur le sens de de leur travail au sein d'entreprises va tout à fait dans le bon sens maintenant si j'étais taquin, je dirais que pour la qualité du débat, il est important qu'on ait les meilleures données et que la qualité donc des publications extra-financière que vous avez refusé tout à l'heure aurait parfaitement permis de mieux éclairer le débat au sein de l'entreprise, donc là je trouve qu'on n'est pas encore totalement en cohérence, mais effectivement cette proposition qui vient de la Convention citoyenne va évidemment culturellement dans le bon sens. Qui vote contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 693 monsieur. si madame la présidente, madame la ministre, notre groupe vient de voter votre amendement, madame la ministre. Mais nous avons nous proposer, donné un avis favorable, juste quand même pour vous dire sur la création sur la création du CSE ça pose beaucoup de problèmes pour les salariés. Parce qu'ils ont beaucoup de questions à s'occuper. Et peu en réalité de temps pour s'occuper des vrais dossiers par exemple quand vous discutez, mais dans le réel, pas dans l'abstrait qu'on discute dans le réel avec les salariés, ce qui était l'ancien Chsct aujourd'hui, les questions de santé au travail, ils ont pas le temps de les traiter, c'est ça la réalité. Et dans beaucoup d'entreprises, écoutez bien, Madame la Ministre, dans beaucoup d'entreprises. Si vous pouvez faire remonter sa Madame Borne, peut-être que vous écoutera donc nous nous sommes partisans de donner une nouvelle compétence sur les questions environnementales, mais vous allez bien voir la patte du groupe communiste républicain et citoyen écologiste, donner un peu plus de temps aussi pour pouvoir exercer cette mission donc pour les entreprises de 50 salariés plus 2 heures et pour celles de plus de 300 salariés 4 heures de délégation supplémentaires, ça ne sera pas de trop pour s'occuper de cette question spécifique environnemental et traité sur les questions de métiers notamment de formation pour les salariés, je vous remercie. Merci, cher collègue, le 1500 22 Monsieur Yates. Monsieur

salariés, selon que l'entreprise est assujetti ou non à l'obligation de négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et parcours professionnels donc cet amendement propose que les représentants des salariés bénéficient d'un surcroît d'heures de délégation. Merci, cher collègue, monsieur le rapporteur, votre avis sur ces deux amendements si vous merci. il n'y a donc pas lieu d'augmenter le nombre d'heures de délégation des représentants du personnel et donc c'est un avis défavorable pour les 2 amendements le 693 et le 1522. Merci, monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. Même avis à partir du moment où l'amendement gouvernemental n'a pas rétabli la rédaction initiale par souci de cohérence, donc je j'émets un avis défavorable. Merci, je mets donc aux voix l'amendement numéro 693 avec 2 avis défavorables qui vote pour.

cet amendement vide vise à favoriser le développement de la sobriété numérique au même titre que la transition écologique : les enjeux liés au numérique et ses conséquences sur l'environnement ne sont pas négligeables dans une société transformée par la pandémie avec notamment un recours plus important au télétravail, il semble opportun d'inscrire dans la loi la nécessité de lutter contre les impacts en face n'efface pardon du numérique sur notre environnement cet cet amendement prévoit donc d'introduire explicitement que cet enjeu du présent, mais surtout de demain doit être pleinement pris en compte dans le secteur de l'emploi.

avec d'autres amendements puisqu'il s'agit du CSA et de la délégation mais bon, au préalable, je dirais sur le la CSA, moi aussi je vais demander 2 heures de de plus par par par mois pour pour s'occuper de de cette mission environnementale et que si on veut décharger le le CSA, il est urgent de rétablir le Chsct hein, il suffit de de regarder toute l'évolution de la santé au travail

qu'y compris dans l'activité économique impose que la démocratie en entreprise prenne en compte la dimension de la transition écologique et les importants changements qu'elle qu'elle cet amendement a donc pour objet de modifier le code du travail pour permettre aux partenaires sociaux dans les entreprises de s'emparer des enjeux de la transition écologique, les salariés dans l'entreprise, ont un rôle à jouer un rôle essentiel pour porter les exigences de la transition écologique au plus près de la production de la machine productive, il vise à doter donc le comité social et économique d'un rôle dans l'adaptation de l'entreprise à la transition écologique et aux conséquences environnementales de son activité, il prévoit au sein du CSA, des entreprises de plus de 5 50 salariés la mise en place d'une commission dédiée, c'est peut-être la différence avec mes 2 collègues une commission dédiée et en conséquence, l'attribution de 2 heures mensuelles de délégation aux représentants du personnel en charge de ces questions à la manque, stage de formation spécifique autour des enjeux d'adaptation des entreprises et des métiers aux objectifs de la transition écologique, il faut mettre la démocratie sociale au service de la transition écologique, c'est une attente des Français et des Françaises et des salariés.

L'amendement 200 soit. 113 présenté par Monsieur Billac. Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le présent amendement outre rétablissement des dispositions de l'article 16 supprimé en commission précise que parmi les sujets sur lesquels le comité social et économique est informé consulter figurent les implications de la transition écologique sur le volume ou la structure des effectifs, il précise également que le CHUV consulté sur les implications de la transition écologique sur la politique sociale de l'entreprise et les conditions de travail et d'emploi. Chers collègues, le 1515 présenté par notre collègue Madame Jourdain. Merci madame la présidente, bon, cet amendement porte évidemment sur l'article 16 Dante nous précédents compte que mais ils ciblent davantage l'adaptation des emplois et des conditions de travail aux enjeux de la tradition et de la transition écologique afin qu'elle soit un sujet de négociations collectives dans le corps de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'objectif poursuivi est d'anticiper les effets de la transition écologique sur l'évolution de la structure des emplois et sur les besoins de formation futur des salariés un autre sens, il est indispensable que ce sujet de négociation soit débattue au sein de l'entreprise, parce que les enjeux de cette transition donc écologiques sont fondamentaux pour l'adaptation tant des salariés que de l'entreprise, donc au futur, la plupart des dispositions prévues à cet article a été supprimé dans le cadre des travaux de la commission notre amendement propose donc de les réintégrer au projet de loi et il propose également de les compléter les conséquences environnementales de l'activité, le entreprises les effets de la transition écologique sur sa situation économique, ces orientations stratégiques doivent en effet faire l'objet d'une consultation récurrente et spécifique du comité social et économique, afin que ces sujets ne soient pas dilué parmi les autres consultations dudit comité. Merci, cher collègue, le 1752 présenté par Madame Havis. Cet amendement vise à préciser que le comité social et économique et consulté sur les implications de la transition écologique sur la politique sociale de l'entreprise et les conditions de travail et l'emploi.

J'aimerais introduire cet amendement par l'évocation de l'histoire professionnelle de Karim Ben Ali Karim Ben Ali est un chauffeur routier employé par Suez Environnement mais en sous-traitance pour ArcelorMittal à Florange, fin 2016, ses employeurs lui ordonne de transporter des matières liquides pour les déverser en pleine nature, il a été contraint de déverser tous les jours, de décembre 2016 à février 2017 près de 28 m3 cube d'un liquide jaune fluorescent ultra toxique, je le cite, à mesure que le liquide s'écoulait sur le sol des rochers éclatés tout autour du lieu de déversement, il y avait des marcassins crevé et lapins qui gisaient au sol et tout un tas d'autres carcasses à même pas de kilomètres d'habitations, j'ai alors décidé de tourner des vidéos, histoire d'avoir des preuves, puis j'ai tenté de faire un signalement auprès de mon employeur, mais personne n'a relayé mon signalement au lieu de ça, j'ai été licenciée à cause des produits toxiques je transportait, j'ai eu une perte de goût et de l'odorat et des irritations au niveau des yeux maintenant je vis aurait RSA c'est ça, ma vie est foutue, aujourd'hui l'histoire de Karim Ben Ali et celle d'un lanceur d'alerte qui a été contraint de réaliser un acte illégal et polluants, sans qu'aucun dispositif au sein de l'entreprise n'ait pu être activé et sans que la législation n'est plus lui conférer une protection nécessaire au moins le temps de l'instruction du dossier, l'objet de cet amendement et donc de renforcer le dialogue social en entreprise, en accord avec les objectifs écologiques de ce texte, il s'agit d'élargir les compétences du cesse en lui attribuant un droit de regard sur les orientations de l'entreprise en matière de lutte contre le changement climatique, tout en instaurant un droit d'alerte écologique en continuité du droit d'alerte sociale qui existe déjà, afin de mettre en place des procédures adaptées à l'étude de ce genre de dossier au sein de l'entreprise et protéger les employées qui défendrait l'intérêt général en alertant les autorités. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur, votre avis sur ces six amendements. La sobriété numérique n'a pas de lien évident avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, elle ne devrait pas relever de la régulation de branches, au demeurant, on peut considérer que ce thème constitue un aspect de la transition écologique et donc pour cet amendement à 49, ce sera une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable sur les 5 autres amendements, c'est un peu le même argumentaire que j'ai pu développer la s'il y a, il y a quelques minutes sur le fond, les comités sociaux économiques viennent d'être mises en place suite à à une des ordonnances de 2 septembre 2017 ils sont prématurées d'élargir leur mission alors qu'ils peinent encore à se saisir de la plénitude de leurs attributions en outre les réformes récentes ont cherché à laisser davantage les acteurs de l'entreprise définir leur agenda en levant des contraintes juridiques, conduisant à des consultations uniquement formelle ces amendements vont à l'encontre de cette dynamique que l'on retrouve au sein des des entreprises et donc il est proposé d'émettre un avis défavorable aux amendements 853 273515 1752 et 423. Merci, monsieur le rapporteur, Madame la Ministre votre avis. du numérique, ils sont déjà tout à fait induit dans la notion de prise en compte des enjeux liés à la transition écologique qui est mentionné à la. Le 16 qui prévoit bien que les négociations collectives au niveau de la branche comme des entreprises en matière de gestion prévisionnelle des emplois, des compétences devront tenir de c'est ne tenir compte de ces enjeux, donc c'est une demande de retrait car satisfait, sinon avis défavorable sur les autres amendements sur ce proposant le rétablissement dans un 1er temps de la rédaction, sorti de l'Assemblée nationale, de l'article 16, évidemment que le sentiment est favorable, par contre ils intègrent tout ça un renforcement d'attribution nouvelles du CSE, qui me semble alourdir exagérément le le fonctionnement du CSE et puis à ceux qui prévoit l'intégration de ces considérations de transition écologique mais en silo, si j'ose dire, je n'y suis pas non plus favorable dans le sens où je pense que ces considérations, elles doivent être partie intégrante de toute réflexion et de tous les travaux et pas étudié ponctuellement et et en silo, ce sont donc des avis défavorable sur les amendements de 173000 515752 423 et 853. Merci madame la ministre, l'amendement 49 et retirée ou vous le maintenez Monsieur boulons. Retiré merci. Je mets donc aux voix l'amendement 853 avec 2 avis défavorables qui vote pour. Abstention : il n'est pas adopté ce que je peux considérer que c'est le même vote sur l'ensemble des amendements même vote, ils ne sont pas adopté 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune 272. Monsieur Guillaume. afin qu'ils proposent des actions concrètes sur les mutations professionnelles liées aux filières, et au mythe aux métiers de la transition écologique et énergétique à vue de nourrir les négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, je vous remercie. Merci, cher collègue, l'amendement 1670 présenté. Oui, madame la présidente, c'est un amendement très proche du précédent, l'article 16 de ce projet de loi renforce la prise en compte des enjeux de la transition écologique dans les négociations de branches et professionnel et à cette fin, l'amendement renforce le rôle des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications afin qu'ils proposent des actions concrètes sur les mutations professionnelles liées aux filières et aux métiers de la transition écologique, l'objectif étant de rendent plus opérationnels, les négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Merci madame filiale votre avis, monsieur le rapporteur sur ces deux amendements s'il vous plaît, merci. Si madame la présidente, ces amendements ont déjà été présentés en commission, le rôle d'un observatoire, et en l'espèce, l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications n'est pas de formuler des propositions si les branches identifie des propositions concrètes, rien ne les empêche de les formuler, en revanche, si elles n'ont elles non n'identifie pas, excusez-moi, il n'est pas pertinent de les obliger par la loi, le faire il est proposé un avis défavorable sur ces deux amendements 272 rectifié et 1000 600 70. Merci, monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. ces amendements, il vise à renforcer le rôle des observatoires donc dans cette négociation, en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau de la branche qui est prévu par l'article L 22 41 12 qui s'appuie sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, il précise que cet observatoire, il porte une attention il porte une attention particulière aux mutations professionnelles et il le complète les missions confiées aux observatoires en prévoyant qui. Propose des actions concrètes quant aux mutations professionnelles liées à la transition écologique alors effectivement cela alourdit un petit peu l'émission de ces observatoires mais cette proposition, je crois qu'elle pourrait permettre aux observatoires de faire des recommandations d'actions concrètes en matière de VPC aux commissions paritaires nationales de l'emploi, les instances politiques des branches professionnelles, c'est donc un avis de sagesse avec un un sentiment très favorable. Merci, je mets donc on voit cet amendement 1876 avec un avis défavorable de la commission très favorable du gouvernement qui vote pour. Qui vote contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté même vote pour le 1670. Même vote il n'est pas adopté, je mais on voit l'article 16 qui vote pour. Contre, abstention il être adopté une façon maintenant à l'article 16 avec un amendement du gouvernement, le numéro 21 53 Madame la ministre. Merci madame la présidente, économiques et sociales en base de données économiques, sociales et environnementales, ainsi que l'obligation d'inclure dans cette base des informations qui soient relatives aux conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise, il rétablit ensuite le texte qui prévoyait d'élargir la mission de l'expert comptable intervenant en tant que conseil du comité social et économique à l'appréciation des conséquences environnementales de l'activité de l'entrepôt les modifications qui ont été proposées en commission au Sénat qui supprime l'ensemble de ces dispositions, elle prive le comité social économique d'un rôle prépondérant, je crois, en matière de transition écologique et donc cette proposition s'inscrit en parfaite cohérence je crois avec avec les dispositions adoptées précédemment. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis cet amendement du gouvernement. Madame la présidente, la commission a supprimé les dispositions relatives à la base de données économiques et sociales et au rôle de l'expert comptable en matière environnementale concernant la base de données économiques et sociales, elle semble aujourd'hui peu utilisé par les élus au CSE, alors même qu'elle représente un travail important de compilation parler pour les entreprises. Cet article imposerait à l'entreprise de mettre à disposition des informations sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise, dont elle ne disposent pas nécessairement et qui peuvent être difficiles à obtenir la contrainte sans le donc excessive, surtout pour les petites entreprises concernant la saisine de l'expert- comptable par le CSE, ce dispositif est peu opportun dans la mesure où les experts comptables à priori ne sont pas les professionnels les plus à même d'apporter au CSE, des éléments d'ordre environnemental, de nature à améliorer sa compréhension des orientations stratégiques des comptes et de la politique sociale de l'entreprise, en conséquence, il est proposé un avis défavorable. Merci, je mets donc aux voix cet amendement du gouvernement avec un avis défavorable de la commission qui votre tour. Contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 1516 monsieur Houlgate. Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, donc, cet amendement, donc, a pour objectif de 2 permettent justement aux représentants des salariés de mieux s'approprier au sein du comité social, économique, les enjeux de la transition écologique et c'est pour ça que nous proposons de compléter donc la base de données économiques, sociales et environnementales par des éléments qui concernent les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise, le bilan de gaz à effet de serre, tels que définis, l'article L 229 25 du code de l'environnement. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît. Alors c'est un avis qui va être très rapide pour les, pour les mêmes raisons évoquées à l'instant, à l'occasion de de l'amendement déposé par le gouvernement, c'est un amendement revient sur la position établie en commission et donc c'est un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Sur le 1er volet vous aurez compris que j'aurais pu être largement favorable sur le second, par contre, il me semble qu'il est satisfait ces données : un sur le bilan d'émissions prévues au Code de l'environnement, elles sont en effet déjà disponible sur la plateforme publique de l'Ademe, c'est donc une demande de retrait.

Abstention : il n'est pas adopté, je mais aux voix, l'article 16 bis qui vote pour. Contre, abstention il être adopté l'amendement 1517 Monsieur Houlgate.

pour maîtriser les enjeux de la transition écologique et se préparer à l'utilisation des informations environnementales dans le cadre des informations consultation et de la gestion des emplois et parcours professionnels, le besoin d'une montée en compétence des partenaires sociaux dans l'entreprise, sur ces sujets et donc essentiel pour engager un véritable dialogue économique, social et écologique. Cette amende demain propose ainsi d'ouvrir aux élus du comité social et économique et aux délégués syndicaux au cours de la première moitié de leur mandat, une journée de formation obligatoire, soit 7 heures pour pouvoir se former aux enjeux environnementaux de l'entreprise. Chers collègues, monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente, avis défavorable à cet amendement pour les mêmes raisons que précédemment évoquées à l'article 16.

d'une formation en santé, sécurité et conditions du travail, ils peuvent en outre bénéficier d'un congé de formation. économique, sociale et syndicale et comme évoqué précédemment, me semble souhaitable que la question de la transition écologique, elle intègre toutes ces formations et toutes ces réflexions et qu'elle ne soient pas traités en silo, c'est donc un avis défaveur.

rétablir le texte qu'il avait été élaboré par l'Assemblée nationale et puis un certain nombre d'amendements complémentaires, je dois vous faire part de ma déception, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une guerre de tranchées, alors qu'en réalité, hé bien non, le CSE est vraiment un atout au service de l'entreprise, donc il faut renforcer ses compétences, il faut faire confiance aux salariés à la Europe et à leurs représentants pour justement faire ensemble que dans le cas de la négociation de la discussion du dialogue social et puis c'est avoir une convergence d'objectifs et et de revenir à des choses qui me paraissent moins extrêmement passéiste et et je dirais la la frilosité, voire l'hostilité de de la position de la commission moi me heurte un peu et je pense pas que ça aille dans le sens de l'histoire et dans le sens d'un d'un développement harmonieux de de notre économie. Merci, chers collègues, je mets aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui vote pour. Contre. Abstention : il n'est pas adopté, nous arrivons à l'article 17 avec une prise de parole de Monsieur Gay. Oui merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous voulions dire quelques mots sur le télétravail et l'honnêteté connu à me dire que, avec mon collègue Michel Canevet, ici présents et Martine Berthet à la délégation aux entreprises, nous menons un rapport sur cette question, mais ça sera une prise de parole de mon groupe qui n'a rien à voir avec les travaux que nous conduisons, mais évidemment, nous avons mené un certain nombre d'auditions sur cette question, 3 choses à vous dire madame la Ministre, la première chose, c'est que tous les métiers n'ont pas été télétravail able beaucoup plus de cadres évidemment que d'ouvriers et d'ouvrières et que nous avons vu, par exemple celles et ceux qui font le ménage par exemple prennent le RER B, le 1er à 5 heures 50 ça a été plus compliqué évidemment pour elles et eux la 2ème chose c'est que lorsqu'on on discute avec les salariés dans des conditions où le télétravail a été plus subie sur cette dernière période évidemment que choisi que tout le monde nous dit nous voulons continuer à télétravailler, mais plutôt de façon hybride. 2 jours ou 3 jours par semaine, par exemple, la dernière étude de l'APEC monde que 8 cadres sur 10 souhaitent continuer à télétravailler mais plutôt non pas en 5 jours sur cinq mais plutôt à en système mixte ou hybrides, comme nous le souhaitons et la dernière chose à dire, c'est que, évidemment, il y a eu une négociation avec les syndicats de salariés. Tous les syndicats n'ont pas signé l'accord interprofessionnel, nous allons avoir une proposition de loi sur la santé au travail qui devrait arriver, je crois, si je me trompe pas, début juillet, ici au Sénat, mais il faut encadrer cette nouvelle question parce que, avant la crise, c'était environ 5 % des salariés qui télétravailler très probablement qu'après cette crise, ce sera beaucoup plus, il y a évidemment du positif, par exemple, concilier une vie personnelle et professionnelle moins se déplacer moins de perte de temps, générateur d'au moins de stress, certains y trouvent un équilibre mais d'autres nous disent aussi au contraire que le télétravail, par exemple, les a isolés que ils ont eu, eux par contre une vieille difficulté à en faire le distinguo entre vie personnelle et vie professionnelle que notamment la question du droit à la déconnexion qui est déjà reconnu dans notre droit depuis 2017 a été plus difficile à tenir que avant la crise et donc je pense que, au mois de juillet, nous devrons avoir tous ces débats, en prenant en compte l'ensemble de ces aspects en tout cas, nous y voyons il faut encadrer, non pas pour l'interdire, mais bien pour que chacun et chacune puisse s'épanouir dans son travail, grand-mère. Parfait adorable favorable, donc j'ai mis aux voix, cet amendement rédactionnel, avec un indice favorable du gouvernement qui vote pour. Contre, abstention il est adopté, le 854 représentée par Madame penser Monge. Merci madame la présidente, cet amendement vise à renforcer. Le cadrage des schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation en matière de planification économique relative à la reconversion professionnelle des secteurs sinistrés par la crise climatique avec la stratégie nationale bas carbone la France renoue avec son excellence en matière de prospective et de construction des politiques publiques sur le long terme, les schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation document cadre de référence des politiques régionales d'aménagement du territoire doivent eux aussi évoluer et accorder une attention particulière au secteur d'emplois qui pourraient être impactés par la crise climatique et la nécessité d'adapter notre économie et notre industrie à la transition écologique, la mobilisation des idées jaune a montré qu'une écologie qui ne prend pas en compte son impact social qui pourrait même aggraver les inégalités sociales ne peuvent pas dès lors avoir une profonde adhésion populaire, la puissance publique dispose d'outils et d'une expertise qui doit mobiliser pour accompagner la reconversion professionnelle, avec un impact social positif. Si chers collègue monsieur le rapporteur. Cet amendement. Permettra aux régions d'accompagner et de soutenir les reconversions professionnelles engendrées par la transition écologique. Amendement pertinent et donc c'est un avis favorable. Merci, monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. la préférence pour un maximum de latitude aux régions dans la définition de leur objet dans ces schémas et donc un avis défavorable. Merci, je mets donc on voit cet amendement avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui vote pour. Qui vote contre qui s'abstient, il est adopté, je mais aux voix, l'article 17 ainsi modifiées qui vote pour. Contre, abstention il est adopté, l'amendement 856 présenté par Madame Poncet mange. Merci madame la présidente, cet amendement inspiré d'une proposition de la Convention citoyenne peu plus le climat est une demande de rapport visant à assurer l'accompagnement des travailleurs qui risquent de perdent leur emploi dans des secteurs affectés par la crise climatique et la transition écologique, les secteurs français des hydrocarbures de l'automobile, de l'aéronautique et du transport routier ont été affectées par la crise, ça n'était sanitaire alors que leurs effectifs était déjà en déclin déjà en décroissance, à la fois en raison des délocalisations, mais également du fait des nécessaires investissements dans les énergies renouvelables dans le monde, la crise climatique menacerait au moins 80 millions d'emplois ce déclin durable et prévisible, doit s'accompagner d'un plan national de reconversion des salariés des sous-traitants, la transition écologique doit transformer en profondeur notre manière de produire les décennies dans les décennies qui viennent, il est temps que la France anticipe cette révolution industrielle pour être capable de se fixer pour demain un horizon social résiliant cette transition peut être une chance pour les Français en matière de reconversion professionnelle et de création d'emplois et ce doit être le rôle de l'État s'il veut voir la France réussir la transition écologique que d'accompagner les travailleurs et travailleuses à travers leur reconversion professionnelle face à la mutation du monde du travail pour assurer une pérennité sociale à la transition, je vous remercie. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur, votre avis. Merci madame la présidente, ce rapport ne permettrait pas de proposer des solutions concrètes pour accompagner les travailleurs concernés par la perte d'emploi dans les secteurs affectés par la crise climatique et la transition écologique, c'est donc en position d'avis défavorables pour l'amendement 856. Merci madame la Ministre. je crains effectivement que cette ce ce rapport il il est un objet qui est extrêmement l'argent et qui, et qui risqueraient de nous faire manquer la cible une cible que nous partageons évidemment celle d'une transition juste qui répondaient aussi à travers nos objectifs énergétiques à nos standards sociaux, nous disposons de multiples instruments juridiques de l'article 182 la loi du 17 août 2015 jusqu'à la la dernière PPE PPE qui donne effectivement des des cadres et des orientations, il n'est même pas possible de citer toutes les initiatives tant il en existe, on pense notamment au plan d'investissement dans les compétences qui a soutenu les démarches prospectives hein de compétence des branches professionnelles et qui a permis le lancement en 2019 de l'engagement de développement de l'emploi et des compétences de la filière électricité la prochaine PPE ce sera l'occasion de faire un arrêt sur image, si j'ose dire du foisonnement des initiatives lancées depuis 2000 et d'en faire un 1er retour sur expérience dans l'intervalle, je ne crois pas souhaitable d'ajouter un énième rapport, c'est donc un avis défavorable. Merci Monsieur Gay pour explication de vote. Merci madame la présidente, je sais qu'il faut aller vite : je ne veux pas retarder le débat mais je trouve que l'amendement proposé par mon collègue écologiste est extrêmement important parce qu'on on va voir si nous amorçons la transition écologique qu'il faut, il faut transformer des métiers et donc moi je suis désolé madame la Ministre, mais je ne sais pas de quel outil nous disposons aujourd'hui pour faire le bilan de ce qu'il faut transformer comme métier et combien de milliers ou de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'emplois ça concerne par exemple il faut réindustrialiser le pays, et si vous nous voulons réussir la transition par Il faut réindustrialiser le pays et donc là il y a des sources de financement, il y a une ONG qui avait dit qu'il y avait un 1000000 d'emplois dans le climat mais pour l'instant, on n'a pas d'études fiables. Donc c'est pour ça, moi je pense que sur le ce projet, au moins, or c'est un amendement d'appel mais d'avoir un bilan de qu'est-ce qui est au nous pourrions transformer et de quoi, nous avons besoin, je pense que ça serait pas anodin et juste, je finis parce que je sais que dans la dernière période, il en a été beaucoup question,

par exemple l'ont nous dit : oui, c'est un projet écologiquement le greenwashing parce que, en réalité, c'est que Total, qui a perçu. Des dizaines et des dizaines de millions d'euros n'a jamais investi un seul Euro dans le pipeline et la laisser se dégrader et maintenant dit aux 700 salariés bon, regardez, on ne peut rien faire mais vous inquiétez pas, on aura un projet écologique oui mais au passage, ces 500 emplois Directs de détruits, et donc là pour le coup, si on avait un bilan réel, on pourrait aussi préparez ou vous voyez l'avenir avec les salariés qui ont été extrêmement mobilisés ces dernières semaines, je vous remercie. Contre, abstention, il n'est pas adopté, nous passons à l'article 18 avec une prise de parole de monsieur Guey. Oui, très rapidement, merci madame la présidente, madame la ministre de la convention climat avait envisagé des mesures de réduction des injustices sociales et de transformation de l'organisation du travail, l'entreprise n'est pas un espace en dehors de la société et le besoin de renforcer la démocratie s'y applique en 1er lieu c'est le sens de nos propositions qui ont malheureusement une nouvelle fois été déclarés recevables, comme la création d'un droit de véto des comités sociaux économiques sur les licenciements et sur les projets portant atteinte à l'emploi, la santé ou l'environnement, trop souvent, la procédure de consultation ne cesse, en cas de plan de sauvegarde de l'emploi se limite à une obligation formelle ne permettant pas aux salariés de contester le projet de leur employeur, alors même que cette décision peut affecter tout un bassin d'emploi ou nuire aux intérêts économiques nationaux ou aux enjeux environnementaux, nous avions proposé que dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les représentants du personnel dispose d'un droit de véto suspensif sur le projet de licenciement collectif pour motif économique engagée par l'employeur, ce droit d'opposition pourrait s'exercer en cas d'dans l'environnement par exemple en cas d'insuffisance de prise en compte des avis et propositions alternatives du CHU en cas d'atteinte aux intérêts stratégiques d'une filière économique et, par exemple, pour finir aussi faire le bilan des aides publiques qui auraient été versés pour sauvegarder l'emploi et qui malheureusement parfois bénéficie aux actionnaires tout en licenciant des salariés : voilà, nous vous remercions. Merci, chers collègues, l'amendement 50 présentée par. Elles Issa cher collègue Monsieur Jeunet pardon. Merci madame la présidente, cet amendement, souhaite que les entreprises soient informés sur les enjeux liés à l'environnement et au développement durable en abordant expressément l'enjeu de sobriété numérique au regard de la situation actuelle qui a été décrite par mon collègue tout à l'heure à l'article 16. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît. Merci madame la présidente, on on peut se demander si la sobriété numérique n'est pas déjà comprise dans la transition écologique, sinon dans la mesure où l'article 18 charge les autres co-les opérateurs de compétences, d'informer les entreprises sur les enjeux du développement durable ne serait pas beaucoup plus contraignant pour eux d'aborder dans ce cadre, le thème de la sobriété numérique vous ai donc proposé d'une demande de retrait sinon avis défavorable. Merci madame la ministre. Je confirme que l'information des entreprises par les opérateurs de de compétences et déjà prévue par l'article 18 du présent projet de loi et qu'il englobe bien les impacts du numérique, il me semble donc que cet amendement est satisfait, c'est un avis défavorable.

Merci madame la présidente, madame la ministre et chers collègues, la transition écologique implique à moyen et long terme des mutations du monde du travail que les entreprises doivent anticiper afin de ne pas laisser les salariés sur le bord du chemin, à ce titre à la formation professionnelle constitue un levier important, cet amendement précise que le rôle des opérateurs de compétences est également d'analyser les besoins de formation professionnelle, les entreprises auxquelles elles apportent un accompagnement dans l'adaptation à la transition écologique. Si cher collègue 2130 Madame avait même argumentation donc défendu merci, monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente, ces 2 amendements ont déjà été présentés en commission sont satisfaits, car la mission d'analyse des besoins en formation professionnelle relève déjà par nature des OPCA et donc proposer un avis défavorable. est tout à fait partagés, effectivement, il est déjà, elle est déjà induite dans l'émission des eaux, donc c'est une demande de retrait sinon avis défavorable.

Le recours au télétravail est un moyen pour les entreprises de faire face aux enjeux liés à l'environnement et au développement durable, le présent amendement propose donc de le faire figurer expressément dans le Champ de la future mission des opérateurs de compétences, d'accompagnement des entreprises face à cet enjeu. Il monsieur le rapporteur. et de qualification professionnelle, c'est donc un avis défavorable. Merci même avis, Madame la Ministre. Je pense que ces impacts du numérique et il ils incluent un ces ces impacts du télétravail, en tout cas, nous considérons que c'est ces considérations sont déjà prises en compte par l'article 18 s'est donc à nouveau une demande de retrait sinon avis du. Retrait. contre, abstention, l'article 18 est adopté, l'amendement 855 présentée par Madame Poncet mange. Merci madame la présidente, cet amendement vise à proposer aux entreprises de consacrer au minimum 10 % de leurs bénéfices à la création d'un fonds consacré à la transformation écologique et sociale de l'entreprise, selon la Commission européenne en 25 ans, les entreprises européennes ont multiplié par 4 la part des revenus dédié à leurs actionnaires aux dépens de l'investissement, de son côté pour la France, Oxfam relève que, depuis 10 ans, un quart des sociétés du CAC 40 a reversé plus de dividendes qu'il n'a fait de de bénéfices, ce qui empêche ces entreprises de réaliser les investissements nécessaires à leur transformation et à la construction de leur résilience et puis ensuite à demander de l'aide publique pour investir, face à la crise environnementale, ce comportement n'est plus à la hauteur n'est pas d'ailleurs à la hauteur de l'enjeu, aujourd'hui plus que jamais, les entreprises doivent faire face à un défi : celui de développer leur activité tout en se donnant les moyens de tendre vers la transition écologique au sein même de leurs structures en interne pour cela des moyens financiers existent, cet amendement propose donc aux entreprises de se consacrer au minimum 10 % de leurs bénéfices à la création d'un fonds dédié spécifiquement la transformation écologique et social de leur entreprise afin de leur permettent d'augmenter l'impact positif de leur activité, de gagner en résidence, les entreprises ont toute leur part à prendre pour relever les défis de notre siècle, pour contribuer à produire mieux, de façon plus respectueuse à l'égard de notre planète et de l'environnement, les grandes sociétés doivent désormais elles aussi prendre leur part dans la préparation de la transition écologique et privilégier l'intérêt général, aux intérêts privés, quelques fois un peu vorace de leurs actionnaires. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis sur le 855. Oui, la proposition d'amendement sur le 855. Semble présenter un un dispositif particulièrement lourd et écoutent et donc c'est un avis défavorable de la commission. Merci madame la ministre ma ma vie. La création de cette contribution, effectivement elle irait à l'encontre, en tout cas elle serait un signal un petit peu contre-intuitif dans notre effort de simplification de la fiscalité des entreprises et des investissements depuis 2017 avec, on le rappelle, la suppression de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés de 3 % à l'introduction du du prélèvement forfaitaire unique et et sans doute inquiéteraient en tout cas, nuirait à l'attractivité de la France à sa capacité de d'attirer de nouveaux investissements comprenant évidemment au 1er chef des investissements durables, le développement du financement privé dans la transition écologique, il s'appuie sur d'autres initiatives comme la nouvelle taxonomie européenne ou le développement de véhicules d'investissement durable au niveau européen, tels que les obligations vertes ou l'éco-Label, c'est donc un avis défavorable. Merci, je mets donc aux voix cet amendement avec Madame forcément. Pour explication de vote. Oui, madame la ministre, je conçois que vous ne soyez pas favorable à cet amendement, mais il ne s'agit pas d'une contribution, il s'agit de ne pas faire un contre-sens quand même pour s'y opposer, il ne s'agit pas d'une contribution d'une fiscalité, il s'agit d'obliger les entreprises celles dont j'ai parlé, qui distribue plus que leurs bénéfices à leurs actionnaires et qui du coup n'investissent pas de dédier en interne 10 à un fond interne pour assurer la transition écologique et sociale, donc voilà, vous pouvez toujours être contre, mais s'il ne s'agit pas d'une taxation d'une fiscalité ou d'une contribution, il s'agit d'une obligation dit d'affecter un peu des bénéfices, il s'agit des bénéfices à la transition écologique et sociale. Merci, je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui vote pour. Contre, abstention, il n'est pas Z opté, nous passons à l'amendement 1716 Madame Filleul. merci madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, la justice sociale est un enjeu majeur de la transition écologique c'est pourquoi notre amendement propose que l'État s'engage aux côtés des entreprises dont les activités vont être modifiés par ce projet de loi climat et résilience, s'il est en effet urgent de verdir notre économie, il est également nécessaire d'accompagner les entreprises dans un changement d'activité afin que celles-ci puissent maintenir et créer de nouveaux emplois, la transition écologique doit s'accompagner de mesures fortes pour le maintien et la création d'emplois nouveaux, en partant des activités existantes, les mesures écologiques doivent être complété d'un volet social afin d'assurer l'accès à l'emploi. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, il s'agit d'un des multiples projets de 2 rapports portant sur des thèmes très proche et donc c'est un avis défavorable de la commission. Merci madame la ministre. dans les négociations collectives en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour donc au niveau des branches et pour les entreprises d'au moins 300 salariés, l'article 18, il confie une nouvelle mission aux opérateurs de compétences pour accompagner les branches et les entreprises dans l'adaptation des emplois et des compétences à cette transition avec par ailleurs de nombreuses autres outils qui permettent déjà d'accompagner les entreprises et les salariés qui sont touchés par ces mutations économiques, c'est donc un avis défavorable. Merci, je mets donc on voit cet amendement avec 2 avis défavorables qui vote pour. Contre, abstention, il n'est pas adopté. Ce sont maintenant à la l'article 18 heures pardon, 2 amendements du gouvernement, Madame la Ministre, 2154 et de 2249. ce 1er amendement il clarifie la situation des salariés de la branche des industries électriques et gazières, dont l'emploi est menacé, on le sait, par la fermeture des. Centrales à charbon pendant qu'ils sont en congé de reclassement, un congé qui précède le congé d'accompagnement spécifique mis en place par l'ordonnance du 29 juillet 2020 dans les 2 cas, la situation du salarié au regard du statut de 1946 est la même et l'amendement vient de rappeler les salariés, les regarder pendant cette période comme étant en position d'activité au sens et pour l'application du statut national des professionnels des industries électriques et gazières telle que mentionnée à l'article 47 de la loi du 8 avril 46 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, en outre, si le salarié malade pendant cette période, alors son allocation est maintenue, je vous propose donc de d'accepter cet amendement qui sécurise le dispositif juridique de l'ordonnance s'agissant des salariés de la branche des industries électriques et gazières. Merci, monsieur le rapporteur. madame présente Madame le Ministre, chers collègues, sur cet amendement 22 49 l'amendement vise à appliquer. C'est là maintenant 21 54 le 1er pardon pardon pardon, non, non, je vous en prie. L'amendement vise à impliquer à l'allocation complémentaire, les mêmes modalités que le congé de reclassement dans le cadre du filet social afférent aux salariés des entreprises exploitant des centrales à charbon, je vous rappelle, c'est un débat qu'on avait largement eu dans la loi climat, cette évolution permet aux salariés de parce qu'ils soient regardés comme en position d'activité l'allocation puisque n'est pas suspendu en cas de congé maternité, congé paternité ou de d'adoption et le versement est maintenu en cas de maladie, cette modification va dans le sens d'une sécurisation de et d'une harmonisation des conditions de mise en oeuvre et des dispositifs sociaux prévus par l'ordonnance et c'est un avis favorable. Merci, je mets donc aux voix cet amendement avec un avis favorable de la commission qui vote pour. Contre, abstention il être adopté votre 2ème amendement madame la manif. avec cet amendement, de nous revenons sur les dispositions qui ont été introduites par l'examen du texte en commission qui aurait pour effet de proroger de manière excessive la durée du congé d'accompagnement spécifique des salariés concernés par la fermeture des centrales l'ordonnance, elle prévoit d'ores et déjà une durée qui est particulièrement longue d'accompagnement qui peut aller au total sur un accompagnement de de 18 à 24 mois dès lors pour proroger encore cette durée qui pourrait au contraire éloigner le salarié d'un d'un retour durable à l'emploi, nous vous proposons de revenir à une durée je dirais qui qui permettent cette dynamique, ce serait in fine défavorable à la fois aux employeurs qui serait tenu de garder dans leur effectif des salariés pour des durées exagérément longue mais aussi aux salariés dont l'objectif est un reclassement professionnel durable et non le maintien prolongé dans un dispositif d'accompagnement social qui est par nature temporaire et puis ce serait très dérogatoire au droit commun, notamment au congé de reclassement, le plus souvent limitée à 12 mois, il serait donc pas cohérent de prévoir encore une prorogation une Merci, monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît. Oui, madame la présidente, la ministre, je suis très surpris par cet amendement. Très surpris parce que. Je n'arrive pas à comprendre que je serais tenté de dire, c'est même un amendement inadmissible du gouvernement qui s'était engagé à appliquer des dispositions du droit commun prévue dans le code du travail, dans le cas de l'étude d'impact annexée au projet de loi précitée. Et ce même gouvernement qui aujourd'hui veut supprimer le cadrage protecteur introduit par notre commission qui n'est autre que la reprise du code du travail. C'est absolument incroyable. On est complètement à l'envers par rapport aux engagements avec qui avait été pris dans la loi climat par rapport aux auditions qui ont été faites, c'est un avis effectivement défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, je mets donc cet amendement on voit avec un avis défavorable de la commission qui vote pour. Contre, abstention, il n'est pas The adopté je mais on voit l'article 18 heures ainsi qui votent pour, contre, abstention il est adopté, Madame la Ministre, mes chers collègues, en accord avec le gouvernement et la commission, je vous propose de poursuivre nos aux travaux jusqu'à minuit et demi, s'il n'y a pas d'observation, il est, il en est ainsi décidé, nous passons à l'article 19 avec 3 prises de parole Jean-Pierre Moga. Merci madame la présidente, madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Je tenais à intervenir sur ce titre en en ce que la la forêt joue un rôle essentiel dans l'atténuation du dérèglement climatique, tandis que ce dernier contribuent à menacer la forêt dans son existence même, je partage la position de la rapporteure Anne Katerine loisirs le projet de loi climat et résilience n'a pas accordé à la forêt, la place centrale qu'elle aurait mérité, seul l'examen d'un service public à l'Assemblée nationale y a permis d'une part, de reconnaître le rôle du puits de carbone des forêts à l'article 19 bis, et d'autre part de favoriser leur adaptation au dérèglement climatique article 19 bis E et F aussi lors de l'examen, dans une commission des articles pour actif à la forêt, la rapporteure a adopté des mesures afin d'optimiser le rôle du puits de carbone des forêts et de renforcer la résilience des forêts notamment en obligeant les petits propriétaires à dira au code de bonnes pratiques sylvicoles à remplir un programme des coupes et travaux qui apporte des garanties plus sérieuse en matière de gestion durable concernant la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, l'examen en commission, a permis à l'article 63 bis de renforcer la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, tout comme à l'article 64, terre de remplacer la demande de rapport par un dispositif ambitieux prévoyant l'obligation pour les entreprises soumises à obligation de réaliser un plat de vider vigilance à l'application de la loi sur le devoir de vigilance, de 2017, d'élaborer des mesures permettant d'identifier et de prévenir la déforestation associés à la production et au transport vers la France de biens et de services importés dans la production, contribue à la déforestation, cette dernière mesure était d'ailleurs une des propositions du groupe de travail alimentation durable et locale commun à la commission d'aménagement du territoire et du développement durable et à la commission des affaires économiques, je vous remercie.

chers collègues, concernant cet article 19 et qui fait partie je dirais du du projet de loi qui vise à protéger les écosystèmes et la diversité biologique garantir et préserver l'ensemble des hydro-système je rappellerai 2 dans le rapport lié à ce projet de loi et concernant l'article 19 il est rappelé qu'en 2016 notre délégation sénatoriale à la prospective avait réalisé aussi une étude intéressante en 2016 sur l'eau en tant que biens précieux inscrire également le grand cycle de l'eau dans la loi évaporation précipitations ruissellement et infiltrations, j'ai été sollicité, je dirais, comme d'autres collègues dont nos départements et territoires respectifs par nos agriculteurs au niveau des organisations syndicales FDSEA Jeunes agriculteurs qui suscite réellement de de grandes inquiétudes quand ça à certaines mesures, et donc je remercie la la commission, je dirais, pour avoir adopté en commission des amendements et justement qui prennent en compte pour l'article 19 des sollicitations pour l'avenir aussi de de l'agriculture et les inquiétudes légitimes. L'article 19 relatif à la définition nouvelle des écosystèmes aquatiques, une rédaction qui permettrait de prendre en compte les besoins en eau des activités humaines qui est aussi une mesure de bon sens pour aussi prendre en compte largement et soutenir nos agriculteurs et nos exploitations agricoles, donc dans ces 2 amendements. Le le 1er amendement vise à prendre en considération dans l'article 19 les besoins des activités humaines dans la gestion des écosystèmes aquatiques et le second de mon nom, qui était vu aussi adopté en commission qu'on ne verra pas en séance mais je soutiens le le repli vise en cohérence rédactionnelles avec la charte de l'environnement permette la coexistence entre les activités humaines et les écosystèmes aquatiques donc défendent réellement les activités et le monde agricole qu'on on tient aussi collectivement à soutenir, je vous remercie. Merci, cher collègue Monsieur Daniel chassant. merci madame la présidente, madame humanisme, mes chers collègues, donc cet article 19 concerne effectivement la gestion de l'eau et donne prépondérance aux enjeux de préservation la restaurer et de la restauration des fonctionnalités des écosystèmes aquatiques, respect des zones humides, protection de la pollution de la ressource d'eau, valorisation de l'eau et je me félicite de la nouvelle rédaction en commission de cet article que grâce à l'amendement de Madame le rapporteur et aussi Franck Menonville que j'avais cosigné, en effet, la prise en compte des besoins des activités humaines me paraît essentiel pour conserver la possibilité de monter des projets de stockage de transferts d'eau pour garder les territoires vivant et contribuer à notre souveraineté alimentaire, ne pas être tributaire pour la diversification des cultures est tributaire d'autres pays, les agriculteurs sont les premiers à souhaiter la préservation des écosystèmes et la diversité biologique, mais il faut aussi conserver une possibilité d'intervention en cas de nécessité la prévention des écosystèmes aquatiques, n'est pas incompatible avec des souks stockage d'colinéaires pour le dialogue, par le dialogue les agriculteurs seront source de solutions pour lutter contre le changement climatique, mais ils ne doivent pas être pénalisés dans leurs projets ou financièrement, donc oui à la préservation, bien sûr, de l'environnement avec un développement durable et avec un développement économique et social dans nos territoires ruraux. Merci, cher collègue, nous passons donc à l'article 19 avec 2 amendements identiques présentés pour le numéro 83 par monsieur Demilly. Merci madame la présidente, cet amendement reprend un peu les les propos qui viennent d'être tenus, l'article 211 1 du code de l'environnement, définit les principes permettant de garantir une gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et de prendre en compte les adaptations nécessaires au changement climatique, il est un des fondements de la politique française de l'eau et vise à concilier la préservation des équilibres naturels avec les usages anthropique de l'eau, eau potable, irrigation irrigation hydroélectricité loisirs etc, il est donc nécessaire que ces principes essentiels équilibrant les usages de l'eau soit rappelés dans le cadre de cet article qui réaffirme l'importance de la politique de préservation des écosystèmes aquatiques. Merci le numéro 246 Monsieur Chassaing. La président, mes chers collègues, donc l'article L 211 1 du code de l'environnement déficit défini des principes permettant de garantir une gestion durable et équilibrée de la ressource en ont, et de prendre en compte les adaptations nécessaires au changement climatique, fondement de la politique française de l'eau, il vise à concilier la préservation des équilibres naturels avec les usages anthropique de l'eau, eau potable, irrigation hydroélectricité loisirs etc, il est donc nécessaire que ces principes essentiels équilibrant les usages de l'eau rappeler dans le cas de cet article qui réaffirme l'importance de la politique de préservation des écosystèmes aquatiques. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis sur ces deux amendements identiques. Merci madame la présidente, le commentaire sera donc identique pour ces 2 amendements identiques en commission, nous avons modifié la rédaction de cet article 19 afin de concilier ça a été rappelé tout à l'heure, le principe de préservation des écosystèmes aquatiques et marins en tenant compte des activités humaines il par coeur, il est par conséquent superflu de rappeler que la préservation des écosystèmes aquatiques doit tenir compte de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et donc il est proposé avis défavorable à ces deux amendements. Merci madame la ministre, ma vie. Pas si simple non non je je souhaiterais si vous permettez, madame la présidente, vous dire un mot sur cette article 19 et notamment ces ces dispositions qui donne et redonne un rôle essentiel aux rivières aux zones humides et plus généralement aux écosystèmes aquatiques dans l'adaptation de nos territoires au changement climatique, je crois que nous avons là, avec cet art. Cycle 19 et et suivant des dispositions qui reconnaissent vraiment dans la loi l'importance du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques et leur interaction le bon déroulement du processus naturel du cycle de l'eau qui doit garantir que nous aurons dans l'avenir de l'eau en qualité et en quantité suffisante pour les différents usages cet ensemble d'articles, il vient soutenir le travail de terrain qui est réalisé au quotidien et voulait représenté ici, les collectivités territoriales, les syndicats de Rivière, les comités de bassin, les fédérations de pêche et l'ensemble des acteurs de du cycle de l'eau, je crois que d'ores et déjà, nous pouvons nous féliciter. De cette, de cette réflexion et de ces, de ces riches échanges sur ces dispositions qui était importante sur ces articles 83 et 246 l'article 210 1 du Code de l'environnement, indique que l'eau fait partie du Patrimoine commun de la nation que sa protection, elle est d'intérêt général, quand le l'article L 211 un détail les principes de la gestion équilibrée de la ressource en eau, en indiquant notamment que la gestion équilibrée, elle doit prendre en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et elle vise à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, ils vise existent déjà donc simultanément dans le code de l'environnement. Sans que l'un ne Vienne empêcher l'application de de l'autre, nous avons donc je crois ici un ajout qui nuirait à l'objectif général de de clarté, de lisibilité du droit, c'est donc un avis défavorable. Merci madame la ministre, monsieur Houpert vous avez demandé la parole pour explication de vote. La présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voterai pour cette ces amendements parce que mon collègue et confrères Chassaing, parler de retour à l'équilibre, il devrait que pendant des années, on a fait des lois sur la gestion de l'eau sur la gestion de nos rivières et on aboutit à une gestion qui est typiquement administrative et il y a un manque d'humains, souvenez-vous, pour ceux qui sont, qu'on peut de la bouteille qui ont été élus depuis quelques années le DDA était apprécié dans tous les départements. Maintenant, il y a un problème, une confrontation entre les élus et l'Agence de la biodiversité, parce que on a empilé les lois, on a empilé des décrets et on a fait des lois et des décrets parce que nos rivières, nos ouvrages ont subi l'usure du temps et la négligence des hommes, donc on a créé des lois pour faire rétablir la conduite dignité écologique, on a effacé des centaines d'ouvrages sur le Bassin de Seine-Normandie, plus de 500 ouvrages ont été effacés. Et la Bourgogne, le seuil de Bourgogne d'où je viens, d'où vient Madame Losier cette système karstique c'était géré par des moines cisterciens, ça a été créé par des moines cisterciens qui ont fait des ouvrages pour retenir l'eau là où il y avait de la Marne on a effacé ses ouvrages et l'eau va dans les systèmes Arctique hé ben dans la terre, donc avant combattait l'inondation maintenant se bat contre l'étiage donc retrouveront d'humains, et je trouve dommage que qu'on parle de ce problème, parce qu'il faut revenir sur des choses simples sur un article 19 et sur 2 amendements, donc je demande à Madame la Ministre, puisque vous êtes à. Un souhait mon souhait et je pense que il est partagé ici pour qu'on revienne. Sur du bon sens qu'on revienne en arrière et qu'on retrouve des administratifs qui sont près de l'élu invités des administratifs qu'on aime, comme on est des bon merci. Merci, chers collègues, je mets donc aux voix ces 2 amendements avec 2 avis défavorables qui vote pour.

Oui, nous sommes donc sur un un débat important et sans être trop long en introduction, peut-être se dire néanmoins que je ne suis pas sûr qu'autant des mois nous étions avec ces évolutions climatiques ces évolutions de pluviométrie ces sécheresses et inondations et que nous sommes dans l'obligation, nous sommes dans l'obligation d'inventer de nouveaux systèmes de régulation de l'eau et que quand on on en discute avec d'autres en Europe, nos systèmes de bassins où tous les acteurs sont rassemblés sont quand même des systèmes qui sont regardées avec attention et souvent avec même une certaine admiration parce que l'eau et j'ai été moi-même en charge aussi d'une rivière de gestion de niveau d'eau entre les agriculteurs, les chasseurs, les plaisanciers, l'eau, c'est toujours un équilibre toujours un équilibre entre des volontés et des usages qui si on peuvent être contradictoires et ça peut être rapidement malheureusement extrêmement tendue, je vous propose de supprimer les mots en tenant compte des activités humaines à l'alinéa 2 pourquoi. On est tous d'accord sur le fait de truc qu'il faut trouver des accords des compromis, des dialogues sur l'eau, c'est aussi ce que propose l'article 19 dans le projet de loi initial qui qui évoque dès le départ, les activités humaines, mais cet ajout qui intègre évidemment, ça a été dit avant moi, les inquiétudes du monde agricole déséquilibre en fait de l'Arctique. L'article 19 dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale ne remettait évidemment pas en cause la pluralité des usages ou le droit à l'eau, évidemment, bien au contraire il renforcer ce droit en affirmant, comme préalable, le devoir de protéger cette ressource bien commun en reconnaissant c'est ça en fait de la question importante qui est sur la table ce soir qui est dans l'hémicycle en reconnaissant l'importance des écosystèmes aquatiques comme Patrimoine commun essentiel pour la biodiversité pour les activités même pour l'adaptation au sens moi climatique et l'atténuation de ses effets, il reconnaît donc ce capital comme une ressource vitale pour les habitants et les activités humaines, c'est en oubliant. La protection et la préservation des écosystèmes aquatiques que sont menacés, nos propres usages de l'eau, notamment agricoles, c'est le cas notamment dans la nécessité absolue de protection aujourd'hui des zones humides parce que si on n'a pas des écosystèmes naturels en bon état sur l'eau,

dire : vous avez 2 il dit l'essentiel : merci, monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente, la commission, je le rappelle, une nouvelle fois souhaité préciser que la préservation des écosystèmes aquatiques tiennent compte des activités humaines dans une logique de développement durable, qui assure la conciliation entre la préservation de l'environnement, le développement économique et le progrès social, il n'est donc pas souhaitable de revenir sur cet équilibre ou au fondement même de la charte de l'environnement et notamment de son article 6 et donc c'est un avis défavorable. Merci même avis, Madame la Ministre. le rétablissement du cycle naturel de l'eau, c'est une condition nécessaire et le seul préalable à toute réflexion sur la ressource qui est disponible et en quantité suffisante à l'avenir et pour tous, introduire dès lors et des d'ores et déjà, la notion d'usage c'est maîtres sans doute le souhaitable avant le possible et donc j'ai un avis très favorable sur cet amendement. Sera parfait. Alors j'ai mis aux voix, cet amendement avec un avis Monsieur Chassaing.

non mais attendez, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai pas beaucoup, je me suis pas beaucoup exprimé dans la soirée, parce que vous savez dans dans des territoires ruraux, il y a pas besoin de croissance, elle se fait déjà, on a une diminution dans les territoires d'élevage, une diminution de la course de la consommation de viande donc une des difficultés dans ces territoires avec une diminution des agriculteurs qui vont être obligés de d'avoir des des productions variées pour avoir des productions variées, il faut souvent irriguées et on demande pas ici de bouleverser d'écosystèmes aquatiques, ni l'environnement, on demande simplement de pouvoir faire des retenues colinéaires d'eau de pluie pas ça me paraît pas être une catastrophe donc je, je, je suis content, effectivement, de la position du rapporteur et de la Commission. Merci, chers collègues, je vais donc on voit cet amendement 1083 avec un avis défavorable de la commission favorable du gouvernement qui vote. Qui

et donc comme on assiste là sur les solutions fondées sur la nature, qui ira et présente un axe essentiel de résilience aurait climatiques et je le redis, par rapport à l'intervention précédente, si nous n'avons pas des écosystèmes en bon état, nous n'aurons pas d'eau, nous n'aurons pas d'eau pour les activités humaines, hé ben, donc là c'est bien l'adjectif naturel qui fait le sens de l'article 19 de l'alinéa 2 donc je vous propose de le rajouter, et je ne suis pas plus long, en m'excusant d'avoir été emporté par le Torrent sur mon intervention précédente. Pas de souci, chers collègues, vous êtes rattrapés à celui-ci, merci beaucoup monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente, la commission a souhaité supprimer la la la mention de l'appartenance des écosystèmes aquatiques et marins au Patrimoine naturel de la nation pour lui préférer la notion de Patrimoine de la nation, il convient de rappeler que le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi souligner la faible normativité de cet article, à ce titre, la notion de Patrimoine naturel n'est qu'une formule déclaratoire dont la portée juridique est incertaine et qui n'emporte pas une meilleure protection de ces écosystèmes en conséquence proposé un avis défavorable à cet amendement 1876. Merci madame la ministre. Il me semble que les services rendus par la nature, comme les solutions qu'elle nous offre plus communément appelé aujourd'hui ces solutions fondées sur la nature, elle constitue effectivement un vrai Patrimoine,

je crois que si, si nous pouvons évidemment et nous devons nous prémunir de d'un débat enfermés dans les caricatures les plus les plus faciles et les plus rapides, nous avons en responsabilité à dessiner les solutions de demain, tout en répondant à des situations d'urgence, urgence et changements liés au au dérèglement climatique auquel les agriculteurs, les collectivités font d'ores et déjà face les épisodes de sécheresse ne sont plus ponctuels et ils sont malheureusement beaucoup trop récurrents pour qu'on les considère encore comme des exceptions, donc nous avons je crois en responsabilité à la fois répondre à des situations d'urgence dans des conditions données et à dessiner aujourd'hui cette ce ce chemin d'avenir en réconciliant ses enjeux, ce qui n'exclut pas évidemment les activités humaines mais qui trouve cet équilibre entre les possibles et les souhaitables entre les ressources et ce que nous pouvons en avoir l'usage. sur cet amendement, qui consacre ainsi solutions fondées sur la nature et ce est ce Patrimoine naturel, j'ai un avis très favorable. Merci, je mets donc on voit cet amendement 1876 avec un avis défavorable de la commission très favorable du gouvernement qui vote pour.

mes chers collègues, je vais lever la séance, nous avons examiné 146 amendements au cours de la journée, il en reste 1419 à examiner sur ce texte prochaine séance tout à l'heure, jeudi 17 juin 10 heures 30 pour la suite de l'examen de ce texte, la séance est levée, bonne nuit.